La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 21 décembre 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. M. Gérard Cornu a fait connaître à la présidence qu'il se démettait de son mandat de sénateur d'Eure-et-Loir, à compter du 30 décembre 2018, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral,

la plus cordiale bienvenue. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Monsieur le président, la procédure d'examen simplifié des textes de loi prévoit un vote en séance, mais sans aucun débat ni aucune possibilité d'explication de vote.

correctement dans cette enceinte. Cela montre à quel point les « gilets jaunes » ont raison de se battre pour qu'il y ait plus de démocratie, plus de transparence. Il faut avoir à l'esprit que, dans cette enceinte, les deux groupes de sénateurs les plus importants représentent les trois quarts des

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, le groupe Les Républicains a souhaité qu'il y ait un débat à l'occasion, non pas de la présentation, mais de la réflexion conduite par le Gouvernement sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Je remercie le groupe de m'avoir fait confiance pour porter sa parole. débat par une observation forte, qui explique et qui légitime nos interrogations : la France, en matière d'économie décarbonée,

à la V République, qui nous a équipés en nucléaire et- pourquoi ne pas le dire aussi ? -aux efforts faits avec l'argent du consommateur d'électricité pour diversifier,

Vous avez pris vous-même un décret, monsieur le ministre d'État, et vous avez présenté un dossier assez intéressant sur les préoccupations et les préférences du Gouvernement en ce qui concerne l'évolution de l'énergie. il y a des questions majeures qui n'ont pas été traitées et qui doivent l'être sur le plan politique, c'est-à-dire en faisant le choix de s'appuyer sur le Parlement. Si nous ne voulons pas traiter ces sujets au Parlement, l'actualité nous rappelle qu'ils seront traités dans la rue, dans des conditions de superficialité et de violence qui ne conviennent pas à notre République démocratique. Je retiendrai, pour ma part, quatre angles pour ouvrir ce débat.

? Nous sommes confrontés, et les dernières semaines nous le rappellent, à un problème de trajectoire carbone, qui a fait ressortir la question majeure des inégalités entre nos compatriotes en matière de mobilité. Pour faire simple, ceux qui peuvent accéder aux transports collectifs bénéficient de subventions, quand ceux qui ne peuvent pas y accéder doivent non seulement prendre en charge leur investissement, mais aussi financer par l'achat de carburant le budget public. C'est une injustice, qui est ressentie comme telle.

la faible émission de carbone par habitant dans notre pays tient sans doute à la désindustrialisation, à comparer à la part que l'industrie représente encore, par exemple, en Allemagne. Nous émettons moins de CO2,

accrédite le sentiment que notre politique énergétique défavorise la majorité des Français sur la partie du territoire national à faible densité, compatriotes ressentent la nécessité d'utiliser la voiture, mais où il y avait cependant des activités industrielles, les services se concentrant dans les grandes métropoles.

clairement votre objectif de 50 % d'électricité d'origine nucléaire, dont on ne connaît pas les motifs, d'ailleurs, mais qui est en quelque sorte une vache sacrée sur le chemin de la sérénité et de la paix énergétiques, d'une réussite du

la diversification de l'offre et la fermeture du cycle, à exister sur le plan mondial, vous laissez cet atout français dans l'incertitude et l'expectative. Comme il me reste peu de temps, je citerai,

mais de la dimension du monde. Si nous faisons trop de nucléaire en France, juge-t-on, pourquoi ne pas vendre à l'extérieur ? Si nous faisons trop d'électricité, pourquoi ne pas la vendre en Europe ? En améliorant

en évoquant le problème de la sécurité et de l'indépendance, sur le plan non pas de la guerre- c'est-à-dire tout ou rien -, mais de la manipulation des prix de l'énergie fossile, qui compromet assez régulièrement la perspective d'investissements dans les activités de diversification énergétique. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre d'État, en conclusion, je vous demande si le Gouvernement a l'intention de proposer au Parlement

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Longuet,

comme stratégique au plus haut sommet de l'État, cette PPE, qui est en quelque sorte la stratégie nationale française pour l'énergie pour les dix ans à venir, est fondée sur deux piliers la baisse des consommations d'énergie en général, d'énergies fossiles en particulier ; la diversification de nos modes de production et d'approvisionnement en énergie. C'est notamment une question de sécurité.

: Conseil national de la transition écologique, Conseil supérieur de l'énergie, Comité d'experts pour la transition énergétique, Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Comité du système de distribution publique d'électricité, mais également États voisins de la France. Bien sûr, nous devons piloter en parallèle, dans ce même délai, l'adoption d'une loi Énergie qui révisera la loi de transition énergétique de 2015, notamment sur la date butoir pour l'équilibrage dans la production d'électricité entre le nucléaire et les autres modes de production, que nous avons décidé

votée sur l'initiative du précédent gouvernement. L'objectif, c'est la diversification, l'équilibre, pour ne pas être trop dépendant d'une seule technologie. Cela nous amènera à fermer 14 réacteurs d'ici à 2035, ...

Je tiens à préciser par ailleurs, monsieur le sénateur Longuet, que, contrairement à ce que vous avez dit, c'est non plus la CSPE qui finance le développement des énergies renouvelables, mais bien la taxe carbone. Il était tout à fait logique que, dans une optique de décarbonation des usages, donc de la baisse des consommations fossiles, cette taxe serve à financer le développement des énergies renouvelables en France. Quant au tarif ARENH, dont vous avez parlé, il est stable,

une plus grande coordination européenne pour pouvoir rendre notre mode de production et de distribution plus efficace au regard des objectifs « climat », mais aussi plus sûr du point de vue de l'approvisionnement en électricité. Nous Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.

les outre-mer sont souvent présentés comme les fers de lance de la transition énergétique, car ils regorgeraient de gisements en énergies renouvelables. C'est sûrement la raison pour laquelle la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose qu'il faut « parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030 avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 taille pour les territoires ultramarins, quand on sait qu'ils sont très dépendants des énergies fossiles. En effet, celles-ci représentaient, en 2017, entre 77 % et 94 % du mix électrique des outre-mer, 32 % seulement en Guyane, grâce au barrage hydroélectrique de Petit-Saut. Cependant, les communes de l'intérieur de la Guyane, elles, ne sont pas reliées au réseau et fonctionnent grâce à des groupes électrogènes au diesel. même plus une gageure qu'un défi, quand, en même temps, EDF promeut toujours des projets de centrales thermiques : trois centrales au diesel, d'une capacité de plus de 200 mégawatts, ont ainsi été mises en service entre 2012 et 2014 à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, pour un coût total de 1,5 milliard d'euros. En Guyane, la première PPE prévoit la construction, d'ici à 2023, d'une centrale au fioul de 120 mégawatts pour 500 millions d'euros. Où donc est la cohérence quand l'État s'engage à ce qu'il n'y ait plus d'installations produisant d'électricité à partir d'énergies fossiles d'ici à 2030, mais qu'il continue à les financer ? Où donc est la cohérence de la loi Hulot, qui interdit l'exploitation des hydrocarbures en France, mais ne s'attaque pas à leur utilisation, quand on sait pertinemment que la société moderne n'est pas prête à se passer du pétrole ? Monsieur le ministre d'État, l'interdiction d'exploitation des hydrocarbures en France n'est-elle pas une mesure destinée exclusivement à la Guyane, qui, pour l'heure, est le seul territoire français susceptible d'en détenir ?

Patient, vous avez raison de souligner que les enjeux dans les outre-mer sont quelque peu différents de ceux de la métropole. C'est pourquoi les outre-mer ont fait l'objet, dans la loi de 2015, de programmations pluriannuelles de l'énergie spécifiques à chaque territoire. territoire. Les premières ont été récemment adoptées, donc il y aura un décalage d'environ un an avec la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la métropole. En ce qui concerne la production d'électricité,

de la population. C'est le cas en Guyane. À ce moment-là, la programmation pluriannuelle de l'énergie permet d'assurer la sécurisation de l'approvisionnement en renouvelant des installations,

encore une fois un peu décalées, permettront de mettre la priorité sur la maîtrise de la consommation, mais aussi sur le développement des énergies renouvelables. Nous avons engagé des discussions avec EDF et la Commission de régulation de l'énergie pour voir si, dans le

ont finalement conduit à un alourdissement très net de la facture énergétique des ménages, fragilisant ainsi les plus modestes. Certes, le législateur a qualifié l'électricité de « bien de première nécessité », mais il est impératif, si nous voulons véritablement endiguer la précarité énergétique, de franchir une nouvelle étape et d'appréhender l'énergie comme un bien commun de l'humanité. La lutte contre la précarité énergétique ne doit pas relever des seules politiques sociales. Il faut la placer au coeur de la politique énergétique, les questions de production, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique, que ce soit dans les transports, les logements ou le système productif. C'est aussi cela la transition énergétique : une transition sociétale où l'accès à l'énergie tout au long de l'année devient une nécessité impérieuse pour éviter l'exclusion

par les bouleversements climatiques sont les plus pauvres, alors qu'ils sont les moins responsables de la situation. La seconde visera à indiquer qu'il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale et pas de justice sociale sans transition écologique. Parmi les revendications actuelles, la plus juste et la plus socialement protectrice est la rénovation thermique des logements. Or c'est l'une de nos plus graves carences. D'une façon plus générale, l'efficacité énergétique doit être considérée comme une énergie à part entière. Répétons-le, c'est la plus propre, la moins chère, la moins délocalisable et la plus compétitive. En matière d'économies d'énergie, nous avons là un gisement colossal. Compte-t-on booster les dispositifs d'aides énergétiques, monsieur le ministre d'État ? Compte-t-on favoriser aussi un vrai travail de pédagogie, permettant aux Français de modifier leur comportement en préférant le toujours mieux au toujours plus ? pour parvenir aux 50 % d'électricité nucléaire d'ici à 2035, il faudra tripler l'éolien et quintupler le photovoltaïque. Or, par les demi-mesures que vous venez d'annoncer sur l'éolien flottant, vous risquez de condamner cette filière naissante, en Méditerranée notamment. Dans ces conditions, comment pourrons-nous atteindre les 40 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030 et comment compensera-t-on la baisse du nucléaire en 2035 ? qui peut nous permettre de bâtir une nouvelle industrie décentralisée et porteuse d'un nouveau dynamisme rural, comptez-vous agir pour une simplification réglementaire et pour des tarifs d'achat adaptés ? Très bien ! La parole est à M. le ministre d'État. Monsieur le

Monsieur le ministre d'État, suivant l'avis de RTE du fait des retards de la centrale à gaz de Landivisiau et du nucléaire à Flamanville, le Gouvernement a retardé la fermeture de la centrale de Cordemais, en ouvrant la voie à sa transformation en centrale de valorisation des bois de classe B dans le cadre du procédé Ecocombust. Cette prolongation a évidemment ouvert un débat sur la question de savoir si vous alliez tenir les engagements pris par le Président de la République quant à la sortie du charbon. Première question très simple, monsieur le ministre d'État : cette position sur Cordemais

du site à Landivisiau, de l'abandon possible de ce projet de centrale à gaz qui pourrait devenir inutile en Bretagne

Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, l'hydroélectricité est actuellement la première des énergies renouvelables. Elle joue un rôle primordial pour le système électrique français. Elle représente une production d'environ 10 % de la production électrique nationale, totalement décarbonée et sans production de déchets toxiques. Elle est souple, flexible, permet une grande réactivité, et on estime qu'en hiver, en période de pointe, sur 4 est d'origine hydraulique. C'est en France une filière industrielle d'excellence, dont le savoir-faire s'est bâti historiquement. Alors que, dans le monde, la gestion de l'eau, en particulier pour la production d'énergie, est un enjeu critique de géopolitique, curieusement, le silence entoure en France l'énergie hydroélectrique. On la traite comme une vieille dame respectable ayant vocation à être dépassée. L'objectif de programmation est d'augmenter la capacité de production hydroélectrique de 500 à 750 mégawatts et la production de 2 à 3 à l'horizon 2023. Autant dire une ambition marginale au regard des efforts faits en direction de l'énergie éolienne terrestre. Dans le même temps, nous apprenons que Bruxelles veut imposer l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques EDF. Des dizaines d'ouvrages en France seraient concernées. Aucun autre opérateur européen n'est sommé, comme EDF, de laisser ses barrages ! La sécurité de l'approvisionnement énergétique nationale est une priorité absolue. L'optique qui consiste à privilégier la concurrence pure et dure entre opérateurs met au second plan la politique énergétique. Dans ce contexte, pouvez-vous me dire, monsieur le ministre d'État, quelle est votre position : souhaitez-vous renforcer la filière hydroélectrique en France, augmenter la part qui lui est assignée et en faire un pilier de la transition énergétique nationale ? ? Entendez-vous vous opposer à la privatisation de nos barrages, conservant ainsi dans notre patrimoine national une carte maîtresse de notre indépendance énergétique ? La parole

pas simplement une vieille dame, avec tous les égards que nous lui devons ! Si certains barrages sont plus que centenaires, ils représentent une énergie d'avenir, une énergie propre, qui peut même gagner en efficacité. Il n'a jamais été question de privatisation. Les mots ont un sens. Une privatisation signifierait que l'on vend

n'a été ouverte pour les renouveler, ce qui place nombre de territoires dans une situation d'incertitude que l'on ne peut absolument pas maintenir. Vous le savez aussi, en France, les différents gouvernements ont mené des négociations avec la Commission européenne pour examiner les conditions du renouvellement de ces concessions. Certains voulaient

monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, le Gouvernement a fixé des objectifs ambitieux de transition énergétique dans la programmation pluriannuelle Se doter d'objectifs forts n'est pas nécessairement un exercice difficile. Ce qui est plus compliqué, c'est de les atteindre, et de les atteindre vite, car 2030, c'est demain. La Commission européenne a, en novembre dernier, adopté une vision stratégique afin de parvenir à une économie prospère et neutre pour le climat d'ici à 2050. Le captage et le stockage du carbone sont l'un des sept axes de travail pour atteindre la neutralité carbone. À juste titre, car, selon l'Agence internationale de l'énergie, le stockage de carbone serait le troisième levier le plus efficace pour assurer la transition énergétique. Pour réussir à limiter la hausse des températures mondiales à 2 degrés à l'horizon 2060, il faudra que 14 % des réductions cumulées d'émissions proviennent du captage et du stockage de carbone. Emprisonner et enfouir le carbone émis avant son émission dans l'atmosphère, principalement dans les centrales électriques et les sites industriels à forte intensité énergétique, est essentiel. Si ces technologies sont testées avec succès, elles restent limitées à quelques sites dans le monde et ne sont pas du tout attractives au niveau financier, ce qui bride leur multiplication. À ce jour, le volume d'émissions traité par 18 grandes installations dans le monde est de 40 millions de tonnes par an, alors que l'objectif fixé pour 2050 est d'environ 10 milliards de tonnes de CO2 par an, soit 250 pouvez-vous nous dire où en est la France dans le développement des technologies innovantes de captage et de stockage de carbone ? Nous avons la chance, en France, de posséder un grand établissement public, le Bureau de recherches géologiques et minières, plus communément dénommé BRGM. Ses recherches et ses travaux sont-ils utilisés à leur juste valeur ? Qu'en est-il du projet européen

poursuivre dans cette voie et suivre de près la réalisation de ce projet, qui permettra peut-être d'avoir de meilleurs résultats que les précédentes expérimentations.

semaine prochaine, alors que le Président de la République lance aujourd'hui même le grand débat national. Première question : la PPE pourra-t-elle être revue en fonction des résultats du grand débat national ? Je n'ai pas besoin de rappeler qu'à l'origine du mouvement il y avait la taxe carbone. Le Gouvernement avait élaboré son projet de PPE en fonction de la trajectoire carbone prévue. La suspension des hausses finalement décidée ne vous oblige-t-elle pas à revoir votre copie ? Je pense, par exemple, au soutien aux énergies renouvelables thermiques, dont le niveau dépend beaucoup de la taxation des énergies fossiles.

Uniper a annoncé être entré en négociation exclusive avec un groupe énergétique tchèque pour la vente de ses actifs. Comment réagissez-vous à cette annonce ?

question claire, réponse claire : le grand débat n'a pas vocation à tout remettre en cause. Nous avons pris un certain nombre d'engagements, fait un certain nombre de choix politiques depuis les élections de 2017. Je pense que nous sommes tous d'accord pour considérer que, la légitimité des élections, c'est la légitimité politique par excellence. La programmation pluriannuelle de l'énergie,

situe aujourd'hui au troisième rang des pays de l'Union européenne qui ont la taxe carbone la plus élevée. En ce qui concerne les centrales à charbon, je le redis, notre volonté politique est de les fermer d'ici à 2022. Quatre sites,

qui est en négociation pour racheter Uniper. Cela ne change rien à notre objectif. Quant aux barrages et à l'hydroélectricité, oui, nous considérons que quelques centaines de mégawatts supplémentaires pourraient être valorisées. Tant mieux, mais, vous le savez comme moi, il n'y a pas de grandes capacités pour construire de nouveaux barrages en France. On parle souvent de l'acceptabilité territoriale, citoyenne, sociale, environnementale et économique

En octobre dernier, nous avons reçu ici même M. Jacques Archimbaud, vice-président de la CNDP. Il nous a présenté les conclusions de cette consultation exceptionnelle, qui a mobilisé des milliers de citoyens. Il a insisté sur des points essentiels, dont auraient dû s'inspirer le Président de la République et le Gouvernement pour saisir les attentes sociales et écologiques profondes des Français. Voici, pour mémoire, un extrait de ses propos : « Pour être efficace, une politique énergétique devrait associer mieux les citoyens et les territoires. Largement attachés à donner un plus grand rôle aux collectivités, intéressés par le développement de l'autoconsommation, les participants soulignent que le rôle de l'État doit être de garantir la solidarité entre usagers et entre territoires. Le travail de concertation a donc, d'une certaine façon, déjà eu lieu, monsieur le ministre d'État, mais vous avez manqué de lucidité sur la pertinence des remarques formulées, notamment sur la précarité énergétique, qui touche 7 millions de personnes selon les chiffres de l'Observatoire national dédié Aussi, le montant médian des impayés énergétiques atteint désormais 789 euros, soit quasiment 200 euros de plus qu'il y a dix ans. Ces chiffres étaient connus. Je n'évoquerai pas aujourd'hui nos propositions concrètes en faveur du renforcement de la dimension sociale de la future PPE. Toutes les raisons de la crise actuelle sont rigoureusement consignées dans le rapport de la CNDP : on ne peut faire la transition énergétique contre une partie de la population, ou contre les territoires dont nous sommes ici les représentants. Je crois que vous en avez tardivement pris conscience. C'est pourquoi, alors que s'ouvre aujourd'hui le grand débat, comment le Gouvernement envisage d'y intégrer les réflexions portées lors des débats dont l'organisation a été déléguée, sans ménagement, aux maires.

à reprendre quelques-unes d'entre elles. C'est le voeu que je formule, en espérant que vous saurez redescendre au niveau des territoires et des citoyens, pour lesquels vous avez indiqué qu'il y avait beaucoup d'énergie et de potentialités. La parole est à M. Jean-Paul Prince. Monsieur le Prince. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, le secteur qui émet, à l'heure actuelle, le plus de gaz à effet de serre dans notre pays est, comme chacun sait, celui des transports. transports. Or le transport routier dispose dans ce secteur d'une part modale écrasante, au détriment des moyens de transport alternatifs que sont le train et la navigation fluviale. Ceux-ci sont pourtant plus respectueux de l'environnement. Hélas, ils ne représentaient en 2017 que 11,7 % du fret intérieur. Ces chiffres placent la France parmi les mauvais élèves européens en la matière et montrent une aggravation Face à la dégradation de notre environnement et au défi du réchauffement climatique, il serait très important de changer cet état de fait et de faire preuve de volontarisme en la matière. Le transport routier dans son ensemble a un impact environnemental particulièrement lourd. De plus, ce secteur est particulièrement difficile à réformer ; le contexte actuel nous le rappelle. En revanche, une marge de progrès est possible dans la part modale du fret ferroviaire et fluvial. Le 27 novembre dernier, lors de la présentation des grands Président de la République a fait preuve d'un tel volontarisme, en prenant des engagements forts, en particulier dans le domaine du nucléaire et des énergies renouvelables.

Je suis pleinement conscient que les enjeux auxquels l'État doit répondre dans cette PPE sont nombreux et que ses marges de manoeuvre, notamment financières, sont limitées.

l'État conforte le dispositif de compensation pour assurer la neutralité financière de cette mesure pour SNCF Réseau. Nous sommes précis et concrets : c'est un engagement financier, de même que le maintien d'une aide au transport combiné, visant à favoriser ce mode de transport

craignais de voir revenir des « bonnets rouges » ; M. Darmanin avait à l'époque balayé mes remarques d'un revers de manche. Parce que vous n'avez pas voulu écouter le Sénat, vous avez dû céder à la rue. Sans stratégie gouvernementale claire et partagée, vous naviguez à vue sur un sujet qui est pourtant un enjeu et un défi très important de notre siècle : je veux parler de la transition énergétique. Nous attendons d'ailleurs toujours, monsieur le

: de la position du Gouvernement sur l'électrification de la société française ? Son ambition est-elle toujours de renoncer au modèle de la voiture thermique, au profit de l'électrique, ce qui pose des questions en matière d'aménagement du territoire, d'approvisionnement et de consommation énergétique ? quelle trajectoire financière le Gouvernement a-t-il prévue pour se donner les moyens de ses ambitions, à la suite notamment de la remise en cause de la trajectoire de la taxe carbone ? Quelle efficacité énergétique Comment réduire les consommations ? Quelle montée en charge des énergies propres et renouvelables ? Je pense notamment aux réseaux de chaleur. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous indiquer si le Gouvernement compte mettre en place une feuille de route financière précise, à l'occasion de cette PPE, notamment sur la fiscalité énergétique ? Si tel est le cas, quel calendrier

je pense très honnêtement que, si l'on veut faire gagner l'écologie, ce qui est finalement le sens de la vie, il faut alors tout faire pour associer les territoires et leurs habitants. Or sur ce point, honnêtement, vous avez un déficit abyssal.

de la réduction à 50 % de sa part dans le mix énergétique. Certes, on nous annonce 14 fermetures de réacteur. Il y a pourtant un non-sens aujourd'hui à vanter les mérites de cette énergie, certes décarbonée, tant les risques posés pour la sûreté, la sécurité, l'économie et la santé publique sont avérés. Quel sera le prix à payer pour faire du neuf avec du vieux ? Notre parc est vieillissant : 37 réacteurs atteindront quarante années de fonctionnement à l'horizon 2025. Dois-je rappeler que le risque d'accident n'en est que plus grand ? ? Vous le savez tous : rien n'égale en gravité un accident nucléaire. Sur la sécurité, la sûreté et la gestion des déchets, nous ne pouvons pas pratiquer la langue de bois. Oui, le béton de la cuve des réacteurs devient poreux avec l'âge. Oui, l'émergence d'un nouveau risque sécuritaire, par cyberattaques, mais aussi par attaques physiques, est avérée. Oui, le projet Cigéo reste inabouti, et la gestion des déchets radioactifs qui s'accumulent pose un véritable problème. Oui, le développement de la sous-traitance implique une perte de maîtrise technique de certaines opérations. Oui, enfin, le réchauffement climatique posera problème, en affectant l'approvisionnement des centrales en eau de refroidissement.

Que penser aussi de notre dépendance à l'égard de pays fournisseurs où la menace terroriste est réelle ? Le Niger est confronté aux incessantes attaques de Boko Haram ; à Arlit, le site d'AREVA a déjà été attaqué. l'exploitation des gisements d'uranium a conduit à un désastre sanitaire : la population et l'environnement sont contaminés par la radioactivité. Passera-t-on la situation sous silence, comme cela fut fait en France ? Je ne peux que regretter que le Parlement ne soit pas associé à ces enjeux, dans le cadre d'une loi.

qu'il ne l'était lors de l'adoption de la loi de transition énergétique, en 2015. Nous nous situons dans cette orientation générale, mais nous avons été obligés, par principe de réalité,

Bories. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, permettez-moi de vous faire part de mon étonnement à propos de la programmation pluriannuelle de l'énergie dont nous débattons aujourd'hui. Le 27 novembre dernier, monsieur le ministre d'État, vous présentiez la stratégie française pour l'énergie et le climat. Force est de constater qu'à ce jour, bien que cette présentation ait été faite auprès des Français les médias, la future PPE n'a toujours pas été dévoilée ; sinon, un décret en ce sens aurait été Comment ne pas s'étonner, voire s'alarmer, que la stratégie française pour l'énergie et le climat soit dévoilée alors qu'elle est censée s'appuyer sur un document qui n'existe pas ? Rappelons en effet la portée normative de ce document tant attendu, notamment par les différentes filières de la production électrique. Ce document est censé fixer les objectifs quantitatifs pour les lancements d'appels d'offres adressés aux investisseurs, définir les orientations d'autorisations d'exploitation de nouvelles productions, et proposer les différents scenarii de ce que sera la consommation énergétique des Français en 2023 et en 2028. Je note que, sur les quatre scenarii proposés, seuls deux ont été retenus comme bases de discussion pour le débat public. Voici donc mes questions, monsieur le ministre d'État. Les acteurs du secteur de l'énergie, les décideurs locaux et,, les Français ont montré ces dernières semaines leur désaccord sur les méthodes de concertation et de débat public du Gouvernement ; auront-ils à subir les conséquences de nouvelles volte-face et du retard pris sur le sujet crucial de la PPE ? Pourquoi ne disposent-ils pas d'une trajectoire crédible et transparente, notamment sur le nucléaire, qui nous conduirait vers le respect des engagements de la COP21 ? quel calendrier prévoyez-vous pour présenter la PPE au Parlement, comme le prévoit l'article L. 141-4 du code de l'énergie, et pour publier le décret ?

La lutte contre le réchauffement climatique est au coeur des priorités de la transition énergétique élaborée par le Gouvernement. Pour y parvenir, il faut puiser dans deux sources d'énergie : le renouvelable, bien sûr, mais aussi le nucléaire.

Je rappelle aussi que des pays comme l'Allemagne, le Japon, ou encore les États-Unis, qui ont trop rapidement réduit leur part de nucléaire en faveur des énergies renouvelables, ont constaté une stagnation, voire une augmentation, des émissions de gaz à effet de serre.

on investit pourtant massivement : alors que, parfois, des pales sont à l'arrêt, vous proposez de tripler le parc éolien terrestre. Certes, il est nécessaire de diminuer la part du nucléaire dans le mix énergétique. Mais prenons garde aux fermetures précipitées de réacteurs et veillons au renouvellement du parc nucléaire. Monsieur le ministre d'État, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, le Gouvernement a confirmé son objectif de réduire à 50 % la part du nucléaire au sein du mix énergétique en 2035, ce qui nécessiterait la fermeture de 14 réacteurs. Or la France aura besoin d'un socle

de continuer à investir autant dans les énergies renouvelables électriques, alors que l'impératif climatique nous exhorte à donner une vraie place au nucléaire ?

par la domination du nucléaire dans la production de l'électricité, nous assumons cette diversification, et ce pour une raison simple. Il y a bien un atout économique : il ne faut pas passer à côté de l'essor mondial des énergies renouvelables. Cela concerne des entreprises françaises,

le Président de la République a précisé le 27 novembre dernier ses propositions pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Il a notamment retenu comme priorité la baisse de la consommation d'énergie d'origine fossile- le pétrole, le gaz ou le charbon -et la diversification du énergétique, en mobilisant les énergies renouvelables. Le ministre de l'action et des comptes publics a lui-même déclaré que « la réduction de nos émissions de C02, dont près de 70 % résultent de l'utilisation d'énergies fossiles, passe par une consommation d'énergie plus faible et par des énergies plus vertes ». Or, monsieur le ministre d'État, la politique du Gouvernement n'est pas très lisible en ce domaine. J'en veux pour preuve la non-parution à ce jour du décret relatif à la Le Gouvernement promet sans cesse des dispositions pour favoriser le développement et l'utilisation des biocarburants au moment des lois de finances, mais il n'agit pas fiscalement par la suite, mettant à mal les espérances qu'il suscite. nous votons par conviction et par bon sens, souvent à une très large majorité, des amendements visant à soutenir les biocarburants issus de la production agricole, des filières de l'éthanol et des oléagineux. Hélas, le Gouvernement s'emploie à « détricoter » systématiquement ces mesures à l'Assemblée nationale ! Comment le Gouvernement espère-t-il nous convaincre que les efforts fiscaux doivent porter sur les carburants de seconde génération, qui eux-mêmes n'évinceraient pas les carburants de première génération ? Monsieur le ministre d'État, vous n'ignorez pourtant pas que la seconde génération de biocarburants n'existe pas, ni économiquement ni techniquement C'est justement là toute l'hypocrisie du Gouvernement. Sauvons ce qui peut encore être sauvé, car les biocarburants représentent des milliers d'emplois en France et des débouchés extraordinaires pour l'agriculture. Monsieur le ministre d'État, donnez dès maintenant

la politique de maîtrise de l'énergie et de diversification, l'objectif de carburants liquides devrait être de 432 térawatts-heure en 2028 et l'incorporation de biocarburants de première génération de 7 de l'énergie contenue dans les carburants aux horizons 2023 et 2028. La croissance de la part biosourcée dans les carburants qui ne soient pas fossiles doit se faire non pas avec des biocarburants en concurrence avec la production alimentaire, mais grâce à des biocarburants dits « de deuxième génération » à base de bois, de paille ou d'algues, dont la production et l'utilisation sont encore simplement émergentes en France. La programmation pluriannuelle de l'énergie a bien pour objectif de développer cette part. dans la loi de finances pour 2019- c'est valable pour cette année -, a été voté le déplafonnement de certains sucres de betterave- je n'entre pas dans les détails, mais vous les connaissez à savoir 45 % des sucres présents dans le jus de betterave ayant fait l'objet de deux extractions sucrières. Ce mode de calcul est plus avantageux pour la filière des agrocarburants.

le développement des agrocarburants une incitation à l'incorporation pour les opérateurs qui mettent les carburants à la consommation. Au-delà du plafond existant pour les agrocarburants conventionnels, nous limiterons l'incorporation de biocarburants réalisés à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects sur l'affectation des sols. C'est notamment la question de l'importation d'huile de palme ou de soja, qui, vous le savez, fait toujours l'objet de polémiques quand il s'agit des agrocarburants.

à M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le ministre d'État, je vous ai récemment interrogé sur la sécurité du système électrique. Nous avons eu le plaisir de recevoir en Savoie, vendredi dernier, votre secrétaire d'État. Le hasard a voulu que, la veille, le réseau ait frôlé la défaillance et ait été secouru par les industriels électro-intensifs, ceux-là mêmes que rencontrait votre secrétaire d'État. Or, le jour même, la France actionnait deux centrales à charbon, sans que les mêmes industriels soient activés. Si la PPE s'est fixé l'objectif de cinq gigawatts en 2018, vous le savez, monsieur le ministre Or les industriels pourraient satisfaire la totalité des objectifs avec les conséquences économiques que l'on imagine. Il vous revient, monsieur le ministre d'État, de vous engager en faveur de cette politique volontariste et de démontrer, comme vous l'avez annoncé lors de votre arrivée au ministère, que l'écologie peut se conjuguer avec l'économie. L'autre défi, monsieur le ministre d'État, est aussi celui de la mobilité propre, avec le transport ferroviaire marchandises et sa faible émission de C02. Le Lyon-Turin n'est plus un projet, c'est une réalité, avec 25 kilomètres de galeries déjà creusés sur 110 kilomètres. Il dotera la France d'une infrastructure, à l'instar des trois ouvrages existants entre l'Italie, la Suisse et l'Autriche. Le Président de République et le Premier ministre se sont engagés clairement sur ce grand projet européen. Cependant, ce serait un demi-succès si le transfert modal n'était pas la seconde ambition. La France et la Suisse ont le même volume d'activité avec l'Italie, soit 40 millions de tonnes de marchandises correspondant pour chacun à 3 millions de poids lourds. Or, si la Suisse vient de passer à moins de 1 million de poids lourds sur les routes, la France va dépasser les 3 millions, la moitié dans les vallées de Savoie, avec une augmentation de plus de 196 000 poids lourds en cinq ans. L'autoroute ferroviaire alpine lancée à titre expérimental attend depuis 2009 la décision de la plate-forme de l'Est lyonnais

du maximum de reports modaux, tant pour les passagers que pour les marchandises. Cette infrastructure ferroviaire, au-delà de son caractère franco-italien, est d'intérêt européen et elle est d'ailleurs subventionnée à ce titre.

pèsent lourdement dans le budget de nos concitoyens, en particulier pour les plus fragiles d'entre eux et pour ceux dont les trajets domicile-travail sont les plus importants. Elle l'est aussi, parce que, ne nous y trompons pas, les Français sont bien conscients qu'il nous faut changer de modèle pour limiter le changement climatique et lutter contre la pollution de l'air, même s'il faut bien admettre que la France n'est pas le plus mauvais élève de l'Union européenne ni du monde. Dans le domaine de l'énergie, nous avons donc à traiter deux dimensions, dont on a bien vu, ces derniers mois, qu'elles pouvaient se percuter lorsque les efforts n'étaient pas équitablement répartis. Je veux parler des problèmes de « la fin du mois » et de celui de « la fin du monde », selon l'expression désormais consacrée.

7 à 8 milliards d'euros par an dans les années à venir. Même si les coûts baissent très rapidement et que, pour le même prix, si j'ose dire, nous atteindrons des volumes beaucoup plus significatifs, ce seront toujours plusieurs milliards d'euros qu'il faudra bien trouver quelque part. Or c'est là l'un des grands angles morts de ce projet, Jean-François Husson l'a parfaitement souligné. Pour les financer, monsieur le ministre d'État, vous comptiez sans doute sur les hausses de taxe carbone, mais celles-ci ont été annulées- suspendues, nous dites-vous -et l'essentiel des recettes déjà acquises est mobilisé pour alimenter le budget de l'État et financer d'autres baisses d'impôts ; elles ne pourront donc servir plusieurs fois

Je suis d'ailleurs étonnée, monsieur le ministre d'État, de vous avoir précédemment entendu dire que le débat ne serait pas nécessairement considéré ... Ce que l'on sait en revanche de façon certaine, c'est qu'il faudra bien que quelqu'un soit mis à contribution. Au-delà du mode de financement, les premières remontées des cahiers de doléances ouverts dans certaines mairies font apparaître une forte mobilisation contre les éoliennes. Là aussi, nous sommes au coeur des contradictions qu'il nous faudra surmonter entre, d'un côté, le désir de chacun d'avoir des énergies plus propres, et, et, de l'autre, celui qu'elles ne soient pas installées au bout de son jardin, selon un phénomène bien connu, qui n'épargne en réalité aucune des sources d'énergie- nous pourrions dire la même chose avec la méthanisation. Là aussi, nous aurons à rechercher la juste répartition des efforts, par exemple entre les ruraux, qui auront à vivre avec ces éoliennes, et les urbains, qui ne seront pas concernés, mais qui les réclament,

que dans l'habitat individuel. Nous pourrions multiplier les exemples. Il ne faudrait pas non plus que cette demande d'individualisation croissante permise par les évolutions technologiques- pouvoir produire sa propre énergie verte localement et l'autoconsommer -ne remette en cause les valeurs de solidarité et de péréquation qui fondent notre modèle français, en particulier dans le domaine de la distribution d'énergie. Sans garde-fou, un participant à une opération d'autoconsommation collective pourra décider, un jour, de ne plus contribuer à la solidarité nationale en ne finançant plus le réseau dont il croira pouvoir se dispenser les plus éloignés du réseau paieront alors plus cher, et l'on aboutira à moins de solidarité, là où nos concitoyens en réclament toujours davantage. Monsieur le ministre d'État, prenons garde à tous ces risques. La tâche n'est pas facile, je l'admets, mais je pense que, pour l'accomplir, vous gagneriez certainement à associer encore davantage nos concitoyens- à cet égard, nous verrons ce que donnera le grand débat -, mais aussi les parlementaires. De ce point de vue, je connais votre ouverture personnelle à l'idée d'une véritable loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, mais nous en sommes encore très loin : encore aujourd'hui, nous discutons d'un projet de décret. D'autres progrès en matière de transparence et de contrôle parlementaire pourraient aussi être envisagés : je pense en particulier aux certificats d'économies les C2E, qui sont en réalité une quasi-taxe qui ne dit pas son nom, dont le montant atteindra 9 milliards d'euros sur la période 2018-2020 et qui pèse déjà à la pompe et sur les factures, mais dont aucun des éléments, ou presque, n'est approuvé

Mais, chaque fois que vous voudrez bien associer le Parlement, en particulier le Sénat, nous serons heureux de travailler avec vous, avec pragmatisme et avec pour seule boussole le bien des Français, comme nous en avons, je le crois, fait la démonstration ces dernières années.

les membres du groupe Union Centriste et moi-même avons demandé l'inscription de ce débat sur la gouvernance des grands groupes coopératifs agricoles en raison des dysfonctionnements que connaissent certains d'entre de ces derniers et qui inquiètent autant les adhérents que le monde agricole français. Au-delà de l'actualité, cette inquiétude, que je partage, pose aujourd'hui le problème de l'avenir du modèle coopératif français. Ce modèle

Le tissu coopératif français est d'abord un modèle qui structure fortement l'organisation de la production agricole nationale. Il s'agit d'un modèle solide, d'un modèle d'avenir, d'un modèle défendu par les agriculteurs-coopérateurs, auquel tiennent nombre d'acteurs de la profession.

Ce sont aussi 190 000 salariés et près de 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 40 % du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français. ce modèle est aujourd'hui menacé par certaines pratiques et certaines évolutions, qui ont notamment cours dans les plus grands groupes. Il ne s'agit pas de remettre en cause les principes de concurrence, de marché, d'internationalisation et de développement,

Je commencerai par évoquer la gouvernance. Lors du grand débat coopératif de 2018, il est apparu qu'un tiers des adhérents des coopératives estiment que leur voix n'est pas assez entendue.

problème réside dans la désignation des membres des conseils de surveillance. Le principe « un homme, une voix », qui distingue le système coopératif de tout autre, est bousculé, quand il n'est pas piétiné. Pour exemple, et très concrètement, le conseil de surveillance d'un grand groupe fait aujourd'hui en sorte que le coopérateur d'une section vaut trois coopérateurs d'une autre section, alors que, selon le principe « un homme, une voix », cela devrait être l'inverse.

La transparence reste souvent un voeu pieux. Dans les faits, on déploie beaucoup d'ingéniosité pour se conformer à l'exigence formelle d'information tout en dissimulant l'essentiel.

petit à petit dépossédés de leur outil industriel et commercial et empêchés d'exercer leur légitime pouvoir de décision. La seconde menace est l'internationalisation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement que j'ai évoqué est parfaitement entretenu par l'internationalisation, qui reste malgré tout une marque incontournable de ces grands groupes coopératifs. Il s'agit non pas de contrer de contrer cette dynamique, mais de faire en sorte qu'elle s'inscrive dans le modèle coopératif, qui demeure le modèle protecteur de notre excellence nationale. Trois problèmes

arrive qu'une filiale en Belgique soit en réalité sous le contrôle d'une filiale brésilienne, le tout échappant en totalité au contrôle des administrateurs du groupe coopératif français.

coopératifs et la possibilité de produire des dividendes pour les actionnaires des filiales, ce qui est logique, au détriment des coopérateurs. En outre, la complexité de ces montages en filiales, qui créent une vulnérabilité, ne me semble pas assez anticipée.

Le directoire n'étant pas tenu de transmettre à l'assemblée les éléments comptables précis concernant les résultats de chacune des filiales, seuls les comptes consolidés sont communiqués, ce qui rend l'information nécessaire incompréhensible lors des assemblées générales.

Le législateur, conscient peut-être de l'originalité de notre modèle coopératif, de sa pertinence ou encore de sa vulnérabilité, a mis en place depuis longtemps déjà des outils pour garantir son existence, dont le HCCA. Une telle instance, par les missions qui lui sont expressément dévolues, devrait nous rassurer. Or plusieurs dysfonctionnements ont été récemment relevés. Le président du HCCA lui-même, l'ancien ministre de l'agriculture Henri Nallet, été obligé de demander la démission de l'un de ses membres quand il a enfin été établi que celui-ci était par ailleurs avocat d'un groupe coopératif, ce qui créait un conflit d'intérêts.

Face à ces constats, que pouvons-nous faire ? Pour garantir le fonctionnement des coopératives, qui se structurent autour de valeurs qui sont plus que jamais d'actualité, des évolutions nous semblent nécessaires. Il s'agit d'assurer une meilleure transparence

; d'encadrer la gestion et la gouvernance des filiales en imposant le principe selon lequel la présidence d'une filiale doit être exercée par un administrateur coopérateur du groupe de mieux former les élus des coopératives à la gestion et au contrôle de leurs coopératives ; de conforter le statut des administrateurs, en leur donnant les moyens de remplir leurs missions. Les conséquences des dérives de gouvernance et le passage à une scène internationale non contrôlée pourraient avoir des effets très directs sur nos territoires ruraux, qu'il est de notre devoir de préserver.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'en venir au coeur de mon intervention,

Force est de constater qu'elles sont devenues des actrices incontournables depuis de nombreuses décennies, agissant au coeur des filières agricoles, mais aussi alimentaires, et contribuant à leur structuration. Pourtant, aujourd'hui, nous en conviendrons, les coopératives agricoles sont à la croisée des chemins. D'après un récent sondage, 70 % des agriculteurs considèrent que les regroupements de coopératives ne leur sont plus bénéfiques.

est un acteur incontournable, car il occupe une place prépondérante dans le paysage agricole français. Trois exploitants sur quatre appartiennent à l'une des 2 600 coopératives de notre pays.

ou de croissance externe, lesquelles ont modifié la taille et le champ d'activité de nombre de coopératives, certaines d'entre elles ayant désormais une dimension internationale. Dès lors, comment assurer l'équilibre entre les attentes

pour les groupes coopératifs. Les coopératives agricoles ont tellement prospéré que certaines d'entre elles sont devenues des poids lourds de l'agroalimentaire- quelques-unes seulement, mais leur chiffre d'affaires est important -et ont finalement oublié l'esprit coopératif au profit d'un capitalisme pur et dur. comment ne pas évoquer la crise de gouvernance que traverse la coopérative Tereos depuis juillet dernier ? De nombreux membres critiquent ouvertement la stratégie d'internationalisation et de diversification du groupe, laquelle suscite un grand nombre de mécontentements.

privés. Les partenaires privés, apporteurs de capital, peuvent donc peser lourd dans les décisions. Faut-il d'ailleurs rappeler que c'est sous l'impulsion de l'actionnaire américain de la marque Yoplait, General Mills, que la coopérative laitière Sodiaal a créé au Luxembourg,

Il appartenait à notre assemblée- à nous, parlementaires -de prévoir des modalités de contrôle et des sanctions, afin d'assurer l'application effective de ces dispositions, en veillant à ne pas remettre en cause l'équilibre d'exploitation desdites sociétés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis un coopérateur depuis près de quarante

En tant que vigneron héraultais, je suis fier de rappeler dans cet hémicycle que la coopération viticole est née à Maraussan, commune de l'ouest du département, près de Béziers, en 1901, sous la bannière de « Tous pour chacun, chacun pour tous », et que Jean Jaurès est venu la visiter a rendu hommage à ce regroupement de petits propriétaires, en disant : « Les associés de la Société des Vignerons libres travaillent chacun leur tout petit domaine, mais ils ont commencé par avoir un chai commun, une cave coopérative commune. Mais il ne leur a pas suffi d'organiser la vente. Maintenant que, par une première application de l'association, ils ont vaincu l'esprit de défiance, ils vont plus loin : ils commencent à organiser la production. » Voilà, en quelques phrases précises, l'esprit coopérateur toujours plus loin, car, ensemble, on est plus forts, plus intelligents, et aussi plus audacieux. Depuis lors, la situation a évolué et la tendance s'est inversée : si un adhérent égale toujours une voix, certaines voix pèsent plus que d'autres Alors que, à l'origine, 100 % des coopérateurs étaient des pluriactifs, aujourd'hui, les gros propriétaires représentent 30 % des adhérents et exploitent 70 % des surfaces.

Du poids de chaque cave dépend le pouvoir de certains. On oublie alors, parfois, les valeurs de base de la coopération. L'exemple de la coopérative Tereos, qui a évincé certains de ses administrateurs, montre les dérives possibles d'un tel système quand l'agriculteur perd la main.

Peut-on faire marche arrière et retrouver la fraternité et l'esprit collectif des temps anciens ? Si la personnalité des présidents, leur faculté à coconstruire, est le ciment de leur gouvernance, il me semble nécessaire de repenser la coopération, afin d'assurer une représentation plus réelle L'absence d'obligation d'information et de communication pour le président du conseil de surveillance est une entrave majeure à l'esprit coopératif. Il faut aussi prendre à bras-le-corps la formation des administrateurs et la rendre obligatoire. Compte tenu de la complexification de la législation, mais aussi des évolutions techniques et scientifiques dans le domaine agronomique, il est nécessaire de professionnaliser les membres du conseil d'administration ou,, ceux qui aspirent à faire partie de l'exécutif.

Ainsi s'ébauchent, jusque dans ce monde paysan si morcelé, des formes nouvelles et plus hautes de production et de vie. » Pour ma part, j'espère que ces structures sauront revenir à leurs fondamentaux pour que, aux côtés du germe de solidarité, se développe celui de la démocratie participative.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les coopératives constituent des acteurs majeurs du développement économique. Nées de la volonté des agriculteurs de prendre collectivement en main leur destin, elles ont relevé d'importants défis depuis leur création. Force est de constater que le modèle coopératif rencontre de vifs succès économiques. Ses spécificités en matière de gouvernance, laquelle s'inscrit dans le long terme, en font des entreprises non délocalisables, ancrées dans les territoires. En investissant dans leurs appareils productifs, la recherche et le développement, les coopératives agricoles parviennent à rémunérer leurs adhérents et à effectuer un partage de la valeur plus équilibré. Leur résilience leur permet de mieux résister aux crises, grâce à l'importance de leur capital social et de leurs réserves accumulées, qui leur assurent une réelle capacité de développement. Aujourd'hui, en France, une marque alimentaire sur trois est produite par une coopérative. Face à ces évolutions, la gouvernance des coopératives n'a pas cessé de s'adapter pour répondre aux nouveaux défis. Une évolution majeure tient à la multiplication des opérations de rapprochement ou de croissance externe, lesquelles ont modifié la taille et le champ d'activité de nombre de coopératives. Depuis 1999, les coopératives ont l'obligation de consolider leurs comptes. Elles sont aussi soumises aux contrôles du Haut Conseil de la coopération agricole, le HCCA. Par ailleurs, leurs obligations ont été renforcées en 2014, afin de mieux éclairer les associés sur le fonctionnement de leur groupe. Enfin, plus récemment, l'article 11 de loi ÉGALIM a prévu une réforme par ordonnances de la gouvernance de ces acteurs clés de la chaîne de valeur agricole. Une ordonnance en cours de rédaction fait l'objet d'une concertation. Elle devra reposer sur un équilibre précis entre les attentes des agriculteurs adhérents et les exigences du marché. Les coopératives sont indispensables au développement de notre agriculture. Corrélativement, elles doivent s'adapter. Leur transparence et leur responsabilité doivent être renforcées. Pour y parvenir, différentes pistes sont à étudier. Une première piste consisterait à octroyer au HCCA un champ d'action plus large, afin d'en faire une autorité de contrôle et de régulation. Pour cela, deux éléments sont indispensables : le Haut Conseil doit disposer de ressources supplémentaires, afin de mener des expertises plus poussées, et son conseil d'administration pourrait être ouvert à des personnes qualifiées. de confier au Haut Conseil le soin d'établir une charte de gouvernance des grands groupes coopératifs, dont il contrôlerait la bonne application. charte proposerait notamment des procédures rigoureuses de recrutement des managers et leur évaluation par des cabinets labellisés ; des formations obligatoires des élus du conseil d'administration ; la mise en oeuvre de comités permettant un contrôle renforcé des élus la garantie de la séparation des pouvoirs entre le politique, qui oriente et contrôle, et les managers, qui pilotent et rendent compte de leur action. Une troisième piste consisterait à renforcer le rôle et les moyens du médiateur de la coopération, afin de mieux gérer les situations de conflit ou les crises éventuelles. Certaines coopératives agricoles sont soupçonnées de s'éloigner quelque peu de l'esprit coopératif,

situation a été évoquée précédemment. Néanmoins, les difficultés momentanées d'un groupe coopératif ne doivent pas nous faire oublier que la très grande majorité des entreprises fonctionnent parfaitement bien, et ce quelle que soit leur taille. À mon sens, il faut éviter l'simpliste selon lequel la gouvernance des grands groupes coopératifs s'éloignerait des adhérents, tandis que les petites et moyennes entreprises seraient plus vertueuses. En effet, les grands groupes coopératifs disposent d'un contrôle de gestion rigoureux l'implication et le contrôle des administrateurs y sont souvent plus importants que dans les PME ou les TPE. Les enjeux de filière, de marché et de profil des clients déterminent la taille optimum d'une coopérative. De celle-ci dépendra une organisation de la gouvernance adaptée, décentralisée, par exemple à travers des conseils de section ou de région, des conseils d'usine, ou, pour les filiales, des conseils de surveillance, avec, en leur sein, des administrateurs impliqués et bien formés ; ce point est extrêmement important. Soulignons enfin le rôle essentiel des grands groupes coopératifs. Lors de nombreuses crises, ils ont assuré un soutien financier à leurs adhérents. Pour conclure, sociétés de personnes ancrées dans un territoire mettant en oeuvre une solidarité intergénérationnelle, les coopératives agricoles ont démontré leur remarquable efficacité économique, leur capacité à concilier le local et le global et à construire une économie au service de l'homme, du territoire et du développement durable. Alors même que nous nous sommes penchés, voilà quelques mois, sur la loi ÉGALIM, il ne faut surtout pas décourager l'émergence de coopératives en France. Au contraire, il faut inciter aux regroupements, indispensables à l'amélioration du rapport de force, au profit de nos agriculteurs, alors même que seules

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en préambule, je tiens à remercier notre collègue Pierre Louault d'avoir proposé ce débat sur la gouvernance des grands groupes coopératifs agricoles. En préparant cette intervention, j'ai pu me rendre compte qu'il s'agissait d'un sujet d'actualité, mais aussi d'un sujet sensible, en prise directe avec le quotidien de nos agriculteurs coopérateurs. C'est indéniable : la petite coopérative de village n'existe plus. N'en soyons pas nostalgiques. Sa disparition est la réponse aux évolutions de l'environnement concurrentiel. Face à la mondialisation des marchés, face à la volatilité des prix, face à la mondialisation de la distribution, face à l'augmentation du coût réel du financement, le modèle coopératif a muté en taille, mais aussi en structure. Il a muté vers davantage de concentration. Il a muté vers une intégration plus verticale. Il a muté vers une plus grande diversification des métiers. Il a muté, enfin, vers une plus grande internationalisation. Reconnaissons que si des coopératives agricoles jouent aujourd'hui dans la cour des grands, c'est davantage en raison de leur masse importante que de leur message coopératif. Notons également que la législation a accompagné, particulièrement ces quarante dernières années, ce passage d'une logique paysanne à une logique industrielle et commerciale, puis à une logique financière, en assouplissant le droit. cours de cette mutation, les principes fondateurs du modèle coopératif ont parfois été bousculés. La filialisation, en partenariat avec des entreprises capitalistes, a engendré un nouveau type de sociétés, qu'on ne peut plus définir seulement avec les principes coopératifs classiques. D'ailleurs, dans leur communication, les grands groupes coopératifs évoquent davantage aujourd'hui leur finalité et les valeurs coopératives que les principes ou les règles censées les régir. Présents en amont et en aval de leur marché, les agriculteurs coopérateurs prennent plus de risques aujourd'hui. Pour autant, comme cela a été rappelé à cette tribune, les coopérateurs plébiscitent très largement leur modèle et continuent de le percevoir comme un modèle d'avenir. Tout à fait ! Justement, plaçons-nous du point de vue de l'adhérent. Notre collègue Pierre Louault a cité l'exemple d'un grand groupe du nord de la France que je connais bien. Il ne nous appartient pas, ici, d'en faire le procès, ... Très bien ! ... même si nous pouvons regretter la maladresse de certaines décisions, qui font par ailleurs l'objet de saisines judiciaires. Je me permets néanmoins de rappeler le contexte très difficile dans lequel évolue cette coopérative. Il ne faut pas oublier la fin des quotas betteraviers et la chute du prix du sucre blanc. Néanmoins, la crise de la gouvernance que connaît ce groupe lui permet aussi d'avancer. a pris conscience du déficit de démocratie interne, tout en constatant logiquement que, à 12 000 coopérateurs, l'idée d'une démocratie directe est illusoire. Des commissions thématiques territoriales ont été créées, ainsi qu'une commission des finances. Un audit indépendant a été réalisé afin d'attester la véracité des chiffres. Nous le voyons bien, les agriculteurs coopérateurs, de mieux en mieux formés, de plus en plus informés, d'autant plus exigeants qu'ils vivent une période de crise, demandent une grande transparence de la part de leur structure. Dans le même temps, certains coopérateurs attendent avant tout de leur coopérative le meilleur prix pour leurs produits, quitte à prendre quelques libertés avec les principes traditionnels de la coopération. Pour ma part, j'entends les deux. Je veux croire que l'apport de valeur pour l'usager peut cohabiter avec la valeur pour « l'actionnaire » lorsqu'il y a un partenariat avec le secteur capitalistique. Je veux croire qu'il est possible de tracer une convergence entre un « modèle d'affaires » rendu indispensable par une compétition mondiale exacerbée et un « modèle coopératif qui reste proche et vertueux Contre ce qui pourrait être perçu comme un grand écart, l'idée d'un nouveau paradigme doit s'imposer. D'où doit venir ce renouveau ? Je suis ravi que le Sénat se saisisse de cette question. Le groupe Union Centriste soutient naturellement la proposition de notre collègue Pierre Louault d'une mission d'information sur le sujet, alors que le Gouvernement doit « plancher », en ce moment même, sur le projet d'ordonnance sur le statut des coopératives agricoles qu'il a souhaité intégrer dans la loi Agriculture et alimentation. Je souhaite que le Gouvernement entende, au travers de son ordonnance, les propositions que ne manquera pas de formuler le monde coopératif agricole. Je pense que c'est en cours, très naturellement. Eh oui ! Aidons-le à se poser les bonnes questions.

dans certains groupes, de fusionner en une coopérative unique, en éloignant la gouvernance des territoires ? C'est une question. Pour le dire autrement, comment être un colosse sans pieds d'argile ? Il serait intéressant d'étudier comment ont été provoqués les derniers grands rassemblements, et s'ils ont été soucieux de préserver une gouvernance locale. Je suis persuadé que l'une des forces du réseau coopératif réside dans son enracinement dans les territoires, dont les administrateurs demeurent les garants. Cet enracinement, fruit de notre histoire, est précieux et donne un avantage évident aux groupes qui savent le préserver et l'utiliser. Deuxième question que je souhaite formuler aujourd'hui : comment renforcer le contrôle démocratique de la coopérative et, surtout, de ses filiales de droit commercial On le sait, dès lors que les agriculteurs perdent la main, ils ont tendance à rencontrer des difficultés pour dégager des revenus décents. Ils doivent donc réinvestir les organes de gouvernance, y compris ceux des filiales. Mais comment garantir leur implication quand le système mondialisé impose le recours à des cabinets d'audit anglophones, par exemple ? Il y a, évidemment, un important devoir d'information et un enjeu de formation des coopérateurs. Il y a peut-être également besoin, comme le soulignaient deux responsables coopérateurs dans une récente tribune, d'un « référentiel de gouvernance coopérative détaillé » auquel se rattacher. J'y ajouterai la création de comités d'éthique dans les coopératives de très grande taille. Je voudrais évoquer, ensuite, la capacité qui pourrait être donnée aux coopérateurs de déclencher un audit indépendant sur les résultats de leur coopérative. C'est un droit des salariés aujourd'hui dans les comités d'entreprise. Pourquoi ne pas l'élargir aux coopérateurs dans les très grandes coopératives ? Troisième et dernière interrogation, quelle régulation mettre en place pour adapter les coopératives au monde des affaires sans pour autant contredire les valeurs du modèle coopératif ? ? Je ne l'ai pas encore dit, mais, à titre personnel, je suis évidemment très attaché, comme la plupart d'entre vous sans doute, au modèle coopératif. Toutefois, je me pose légitimement la question : ne faut-il pas le doter d'un gendarme qui puisse agir en toute indépendance et impartialité ? Le Haut Conseil de la coopération agricole pourrait-il se voir affecter des moyens supplémentaires pour assurer cette prérogative, afin d'éviter les écueils dénoncés par notre collègue Pierre Louault en ouverture de ce débat ? Mes chers collègues, vous l'aurez compris, j'appelle de mes voeux une nouvelle gouvernance des coopératives françaises, mais coconstruite avec les intervenants du secteur. Il faut conclure, Pas plus tard qu'hier, la fédération des coopératives a annoncé son intention de présenter en février un guide de gouvernance. J'espère que nous y retrouverons un certain nombre de bonnes pratiques. La parole est à M. Alain

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer la tenue de ce débat, sur un sujet en apparence assez technique, mais qui soulève en réalité de grands enjeux pour le monde agricole français. Les coopératives agricoles sont, en effet, un pilier de l'agriculture française : trois agriculteurs sur quatre appartiennent à au moins une coopérative agricole. Ces structures placent l'homme au centre de leur gouvernance ; elles agissent au coeur des filières agricoles, mais aussi alimentaires, et contribuent à leur structuration et à leurs mutations profondes. Comme l'a montré le congrès de Coop de France qui s'est tenu le 19 décembre dernier, les agriculteurs y sont très attachés et le considèrent comme un modèle pertinent. 77 % des adhérents considèrent que le modèle coopératif répond aux défis de demain. Sur les territoires, ce sont des acteurs incontournables de l'emploi et de la formation. Elles participent à l'innovation agricole, à la valorisation des produits, à l'économie rurale et au rayonnement de la France à l'international. 2 600 coopératives génèrent un chiffre d'affaires de plus de 85 milliards d'euros par an, soit 40 % de l'agroalimentaire français. En Europe, on compte plus de 51 000 coopératives agricoles, soit 9,5 millions de producteurs et 675 000 salariés, dans toutes les filières alimentaires. Elles sont donc aussi un pilier de l'économie française et européenne. Le particularisme des coopératives fait qu'elles sont gouvernées d'une manière démocratique. Principes démocratiques, proximité et dépendance réciproque ont pendant longtemps été les piliers de la gouvernance des coopératives. Ils ont permis de maintenir un engagement fort des agriculteurs. Cependant, au-delà de ce tableau idyllique se cachent des évolutions qui peuvent entraîner certains problèmes de gouvernance. Deux transformations mettent aujourd'hui en tension les piliers de cette gouvernance : l'agrandissement de leur base territoriale et la complexification des enjeux, avec une diversification une internationalisation des activités industrielles et commerciales portées par les coopératives. Elles se sont, pour la plupart, développées dans un environnement marqué par les quotas et les prix garantis. Avec la fin de ces derniers, les coopératives agricoles ont dû s'adapter pour entrer de plain-pied dans la compétitivité. Elles ont souvent fait le choix de la diversification au travers de la création de filiales et l'internationalisation des activités, une adaptation nécessaire pour affronter la concurrence sur des marchés mondialisés, mais qui pose de nouveaux défis. En effet, le lien entre les coopérateurs et leur coopérative s'est distendu et, avec lui, les capacités d'orientation et de contrôle des agriculteurs et de leurs représentants se sont affaiblies. Ces derniers mois, des tensions sont apparues dans certaines grandes coopératives, où des membres demandent un renouvellement de leur gouvernance. Les mesures prévues dans la loi ÉGALIM pour réformer les pratiques de gouvernance des coopératives agricoles arrivent donc au moment opportun pour que celles-ci continuent de jouer un rôle central dans l'agriculture et l'alimentation françaises. Nous serons bien sûr attentifs à ce que les spécificités de ce modèle soient préservées, tout en assurant une plus grande transparence et une plus des instances dirigeantes, en fournissant plus d'informations aux agriculteurs et en promouvant davantage les bonnes pratiques. Les mesures doivent être réalistes pour être efficaces et applicables. Des changements sont nécessaires pour que les coopératives françaises continuent à grandir et à se développer. Les ordonnances prévues d'ici au mois peuvent apporter une partie des réponses pour que les coopératives fassent un saut qualitatif en matière de pratiques de gouvernance, mais c'est aujourd'hui surtout au mouvement coopératif de revisiter ses fondamentaux et de faire des propositions ambitieuses au Gouvernement pour projeter les agriculteurs et l'agriculture française dans les défis du XXI siècle.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a quelques mois, la question de l'organisation des coopératives agricoles a été au coeur de nos débats. Ce sujet est en effet une des mesures clés de la loi ÉGALIM. Nous ne pouvions pas traiter de la question du revenu agricole sans nous pencher sur le système coopératif, compte tenu du poids des coopératives de ce modèle. Si nous n'étions pas forcément tous d'accord sur le véhicule législatif à utiliser, nous savons tous ici, sur ces travées, que cette réforme est amplement justifiée et nécessaire : le modèle de la coopération agricole est en transition. Je ne dirai pas qu'il est en crise, mais nous devons le refonder et le réinventer. La mutation et la modernisation de cet espace coopératif sont indispensables à son avenir. Ce modèle si particulier, où un homme égale une voix, qui représente des valeurs d'entraide, de solidarité et de partage, nous devons le cultiver et le renforcer. Le Gouvernement s'est donné six mois pour proposer une modernisation ambitieuse et efficace de ce mode d'organisation, en concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment Coop de France. Ce sujet particulièrement technique justifie aujourd'hui ce temps d'échange et de dialogue, et je salue l'initiative du groupe Union Centriste. Cette modernisation doit répondre à plusieurs objectifs précis. Le premier des travaux à accomplir, c'est l'amélioration des relations entre les associés coopérateurs et leurs coopératives, c'est-à-dire sur les questions de rémunération, de transparence et de conditions de départ. Aujourd'hui, les associés manquent d'informations sur les relations économiques nouées par leur coopérative. Dans certaines coopératives, il est par ailleurs complexe pour eux d'obtenir des informations sur la mise en réserve des investissements ultérieurs ou sur les résultats des filiales. Pour rénover le système des coopératives agricoles et maintenir le rôle exemplaire des coopératives en matière de contractualisation, il est nécessaire de favoriser l'information de l'associé coopérateur sur sa rémunération et sur la redistribution des gains, ainsi que sur ses conditions de sortie de la coopérative, qui doivent être transparentes et non bloquantes. L'ordonnance instaurera également un mécanisme régulier de contrôle et de sanction garantissant l'exemplarité des pratiques. Le deuxième objectif de cette modernisation est d'adapter aux nouveaux enjeux les règles relatives à la gouvernance, aux missions et à la composition du Haut Conseil de coopération agricole. Institué en 2006 par la loi d'orientation agricole, le Haut Conseil manque de moyens et ses missions essentielles sont insuffisamment connues. Elles gagneraient pourtant à être renforcées. Enfin, le troisième objectif de la réforme des coopératives concerne le médiateur. Après trois années d'existence, seuls six dossiers de médiation lui ont été soumis, Le médiateur de la coopération manque de visibilité auprès des coopérateurs et certains lui reprochent son manque d'indépendance et l'insuffisance des moyens dont il dispose. De plus, l'articulation entre le médiateur de la coopération et le médiateur des relations commerciales n'est pas claire. Face à ce flou, le Gouvernement propose de modifier les conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec les médiateurs des relations commerciales agricoles. Cette modernisation du régime coopératif est essentielle pour assurer sa place dans notre paysage de l'agriculture et de l'alimentation. Les 2 600 coopératives présentes sur notre territoire jouent un rôle essentiel pour notre économie, cela a été dit, avec environ 86 milliards d'euros de chiffres d'affaires, pour nos emplois avec près de 165 000 salariés, mais également pour l'aménagement et la cohésion de nos territoires. Le système coopératif participe à l'évolution et à la dynamique agricole que nous connaissons en de nombreux points du pays. J'aimerais profiter de cette prise de parole pour saluer l'action de Coop de France, qui présentera au printemps un code de gouvernance, afin d'accompagner les coopératives et d'apporter des réponses concrètes aux questions qui sont posées dans les coopératives et par la société. Enfin, je salue l'action du Gouvernement, qui prend le sujet dans sa globalité et qui, fidèle à sa méthode, fait le choix de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Monsieur le ministre, votre prédécesseur annonçait un projet de loi de ratification de l'ordonnance pour le

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat sur la gouvernance des grands groupes coopératifs est tout à fait opportun au moment où le Gouvernement prépare l'ordonnance relative à la coopération agricole que la loi ÉGALIM l'a habilité à prendre, contre l'avis largement majoritaire et transpartisan du Sénat. On sait que ce point a fait dissensus, avec d'autres, lors de la commission mixte paritaire qui n'a pas été conclusive. Nous souhaitions ici pouvoir discuter directement, dans l'écoute de toutes les parties prenantes, du contenu des dispositions envisagées. envisagées. Nos collègues de l'Union Centriste ont demandé l'organisation de ce débat à partir des difficultés que rencontre en ce moment la coopérative Tereos, qui enregistre des déficits records du fait de la fin des quotas sucriers, mais aussi de choix financiers à l'international critiqués en interne. Cette crise a pris une nouvelle ampleur l'été dernier, avec la démission de 70 des 73 conseillers de région et l'exclusion de trois coopérateurs membres du conseil d'administration pour avoir été trop critiques à l'égard de la direction. Ces critiques portaient sur la gouvernance « défaillante », le manque de transparence régnant au sein de la coopérative, ainsi que sur une politique d'internationalisation inefficace. L'article 11 de la loi ÉGALIM habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui concernent directement la gouvernance des coopératives. La première de ces mesures- il y a en a huit -prévoit de renforcer la lisibilité et la transparence des informations contenues dans les documents transmis aux associés coopérateurs par l'organe chargé de l'administration de la société ou adoptés en assemblée générale, notamment le règlement intérieur, le rapport annuel et le document unique récapitulatif. La deuxième prévoit d'améliorer la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs des modalités de détermination du prix et de la répartition des résultats de la coopérative au travers de l'élaboration de documents appropriés. Les six autres mesures concernent moins la gouvernance. La question majeure que pose le cas de Tereos est celle des dérives de certaines grosses coopératives agricoles, notamment au sujet de leur stratégie à l'international, et en conséquence le manque de pouvoir des agriculteurs coopérateurs au sein de celles-ci. Au regard de la diminution sensible, ces dernières années, des exportations agricoles et agroalimentaires françaises, au regard aussi des exigences fortes de la société en matière de qualité sanitaire et d'impact environnemental, la compétitivité du modèle coopératif est un enjeu crucial pour notre pays. Je suis un fervent défenseur de toutes les organisations collectives agricoles permettant d'accroître la valeur pour le producteur et la valeur ajoutée des produits transformés, tout en mutualisant les risques de toutes natures, économiques, sanitaires ou environnementaux. La modernisation de l'agriculture française doit aussi prendre appui sur ses coopératives, petites et grandes. Je trouve qu'il est précieux, dans un contexte national général où la question de la participation et de la redistribution est posée, que le principe démocratique soit au coeur de la gouvernance des coopératives, le principe cardinal étant que chaque associé ou sociétaire dispose, sauf dispositions spéciales, spéciales, d'une voix à l'assemblée générale. Au fil du temps, par nécessité économique autant que par opportunité juridique, la coopération s'est complexifiée et, dans certains cas, opacifiée dans ses montages sociétaires. Les opérations de rapprochement ou de croissance externe ont modifié la taille et le champ d'activité de nombreuses coopératives. Certaines possèdent désormais une dimension internationale. Ces adaptations étaient indispensables pour affronter la concurrence sur les marchés mondialisés. Elles le seront encore demain, mais elles posent de nouveaux défis en termes d'organisation et de gouvernance. Le point de vue de certains associés s'est éloigné dans certains cas, les conséquences des décisions prises ailleurs pouvant avoir des effets positifs ou négatifs très importants sur la coopérative ou l'union de coopératives d'origine, la maison mère. Pour maîtriser et retrouver de la valeur dans l'acte de production, de transformation et de commercialisation, les agriculteurs doivent dans certaines configurations- pas toutes, et c'est heureux -, réinvestir les organes de gouvernance. Ils doivent prendre part à toutes les décisions à caractère stratégique qui conditionnent leur propre rémunération dans le moyen, mais aussi le long terme. Ces principes pourraient trouver une traduction dans l'ordonnance attendue, en prévoyant, monsieur le ministre, un pacte stratégique soumis systématiquement au vote des coopérateurs, un accès facilité des coopérateurs à l'expertise ou à l'audit pour toutes les grandes questions concernant les coûts internes et l'organisation, une implication directe des administrateurs de la maison mère dans la gouvernance des filiales. Monsieur le ministre, dans le contexte de la loi ÉGALIM, quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre par ordonnance pour améliorer la transparence interne et la démocratie des sociétés coopératives si importantes pour la rémunération des coopérateurs et la compétitivité de l'agroalimentaire français ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d'abord, souvenons-nous que les coopératives sont le fruit de l'histoire de l'agriculture française. vieilles de plus de cent ans : c'est à la fin du XIX siècle que les agriculteurs ont décidé de créer les premières coopératives, et ainsi de se regrouper et de faire ensemble ce qu'ils ne pouvaient pas faire seuls. Ce modèle positif et constructif les a conduits à organiser le principe des droits et devoirs de chacun. Cela devrait déjà nous permettre de mener une première réflexion sur la contemporanéité de ce principe, car, aujourd'hui, les droits supplantent souvent les devoirs. N'est-ce pas déjà dans ce principe de base que notre problème réside, dans la perception de la gouvernance de nos grandes coopératives ? N'est-ce pas déjà dans l'exercice trop facile de la critique permanente, sans prendre part objectivement aux informations et aux décisions en tant que simple coopérateur qu'une partie de notre problème réside ? Ce modèle d'entreprise coopérative a aussi conduit les agriculteurs à fixer des principes et des règles. Les principes sont de plusieurs natures : investir ensemble en participant, de façon proportionnelle et égalitaire, au capital social

permettre une bonne valorisation du capital social pour constituer un patrimoine à chaque coopérateur. Nos agriculteurs devraient prendre plus de temps pour recueillir l'ensemble des informations et mener une réflexion collective sur ces principes du mieux faire ensemble.

articles des statuts sont d'une impérieuse nécessité, tel l'article 1, relatif à l'obligation faite à la coopérative de collecter la totalité de la production de son adhérent, partout en France, et l'obligation faite à l'adhérent de livrer à la coopérative la totalité de sa production.

Souvent, j'entends les adhérents parler de « la coopérative » au lieu de « leur coopérative ». Que nos coopérateurs soient acteurs, plutôt que spectateurs

Ces grands groupes coopératifs sont souvent la cible de critiques : ils seraient trop gros, trop industriels, trop agroalimentaires au goût de certains. De mon point de vue, ces critiques ne sont pas fondées. Elles ne sont que l'expression de ceux qui refusent de voir la réalité économique de l'agriculture,

Comment ne pas s'enorgueillir de ces grandes marques qui font la renommée de tout un pays, comme Yoplait, Candia, Béghin-Say et beaucoup d'autres ? Ces grandes coopératives font plus encore.

tous ces éléments, et avec 72 % de coopérateurs reconnaissant que le modèle coopératif répond aux défis de demain, distinguons les questions de gouvernance, donc de pratique, et celles de statut, donc de réglementation. Valorisons ce qui a fait ses preuves ! Valorisons la réussite du difficile pari du collectif face à l'individualisme. Je refuse de croire que les grandes coopératives puissent être les victimes expiatoires d'une société en quête de repères, alors que tout me pousse à penser que le système coopératif est l'exemple même d'une gestion fraternelle, qui fait tant défaut à notre société.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier nos collègues du groupe Union Centriste de nous permettre d'aborder, aujourd'hui, le sujet de la gouvernance des grands groupes coopératifs agricoles. Avant d'évoquer en détail cette problématique, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte s'agissant de la réalité des coopératives et de leur rôle dans les territoires, où elles sont devenues, au fil des années, des acteurs incontournables de développement économique et d'aménagement du territoire. En effet, les principes coopératifs sont communs à toutes les coopératives, indépendamment de leur taille, celles-ci étant le fruit d'une longue tradition, issues de la volonté commune de femmes et d'hommes de structurer leur filière pour répondre aux enjeux économiques, réglementaires et environnementaux. les coopératives agricoles ont étendu leur champ de compétences, de la collecte à la commercialisation, pour déboucher sur la mise en place d'entités de négoce dans le domaine des engrais, des produits « phytos » ou des semences, par exemple. Les coopératives offrent aujourd'hui à leurs adhérents une palette de prestations de services innovants, la mise en place d'outils d'aide à la décision ou de gestion des productions. un champ de compétences techniques en interne très large et très diversifié, qui permet de répondre aux besoins des 2 400 entreprises, dont 13 seulement sont qualifiées de « grands groupes » et 130 d'« intermédiaires ». Le tissu coopératif est donc composé, à 93 ce domaine d'activité, pour avoir travaillé pendant trente ans au sein de la coopérative Alpesud, dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. La mise en oeuvre de la loi ÉGALIM et, plus particulièrement, de l'ordonnance visant à rendre incompatibles l'agrément pour la vente de produits « phytos » et celui pour le conseil n'est pas sans poser de grandes difficultés. En effet, le capital de l'activité conseil ne peut être détenu directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales agréées pour la vente : ni filiale ni holding, par exemple, ne sont possibles. Le conseiller indépendant, qui doit être agréé, ne peut pas percevoir de rémunération directe ou indirecte liée à la production ou à la distribution de produits, à leur application en tant que prestataire ou la vente de matériel d'application. L'agrément est renouvelable annuellement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et s'inscrit dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits « phytos », privilégiant les méthodes alternatives. mes chers collègues, un justificatif de ce conseil devra être présenté pour acheter des produits « phytos », sauf si l'exploitation agricole est certifiée, en sa totalité, selon « un référentiel listé par la voie réglementaire pour ses incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits nombre de questions subsistent. Qu'en est-il du conseil en réapprovisionnement, par exemple ? Où s'arrête le rôle du vendeur, qui peut notamment évoquer la « cible » du produit ? Quel sera le coût du conseil indépendant ? Face aux nombreuses évolutions, la gouvernance coopérative n'a cessé de s'adapter. Mais les dernières évolutions règlementaires provoqueront des changements profonds. Je souhaite, pour ma part, que le débat de ce jour nous permette d'en évaluer les conséquences et d'ajuster certaines dispositions.

Avec un chiffre d'affaires global de 84 milliards d'euros, et dans un monde en pleine mutation, il apparaît essentiel d'améliorer la gouvernance coopérative. C'est aussi une demande des adhérents, puisque 32 % de ceux qui ont répondu au questionnaire de Coop de France considèrent que leur voix n'est pas assez entendue et s'interrogent sur le partage réel du projet de la coopérative. Ce modèle a d'ailleurs vocation à être pérennisé. Ainsi, 77 % des adhérents considèrent que le modèle coopératif répond aux besoins de demain.

les modalités de rémunération par unité de volume des associés coopérateurs à la fin de chaque exercice. Ces modalités sont précisées dans le règlement intérieur, notamment l'information sur les deux clés de distribution du résultat : la part destinée aux associés coopérateurs par rapport à la part restant à la coopérative- c'est tout à fait logique -et la part des dividendes remontés des filiales par rapport aux résultats de celles-ci. Le deuxième sujet, c'est la lisibilité des modalités de sortie de la coopérative, avec, notamment, des informations sur le délai de remboursement des parts sociales.

vous avez été nombre à le dire, ne lui permet pas de remplir cette mission de façon effective. Il est donc proposé de renforcer ses possibilités d'action, en vue d'en faire un conseiller

nécessité de légiférer en la matière. Au-delà des statuts, il faut vérifier la conformité de tous les textes régissant le fonctionnement de la coopérative- règlement intérieur, bulletin d'adhésion, etc. et, surtout, la réalité de son fonctionnement pratique. Ce contrôle existe : il s'agit de la révision. Il sera renforcé, avec la possibilité, pour le HCCA,

et à sa faible visibilité auprès des coopérateurs. Il est donc proposé de modifier les conditions de sa nomination pour assurer toute son indépendance. Le médiateur sera nommé par décret, décret que je prendrai après avis du comité directeur du HCCA. me semble-t-il, que ce soit une personnalité indépendante et que l'on connaisse son existence ! Par ailleurs, l'intervention du médiateur de la coopération agricole doit être mieux coordonnée avec celle du médiateur des relations commerciales agricoles, point sur lequel, effectivement, la marge de progression est assez grande.

Ces priorités sont de renforcer la transparence de la coopérative sur la rémunération des associés coopérateurs et d'assurer le contrôle de cette transparence par le HCCA et le médiateur.

311 jours par an et par coopérative -, on met en évidence le caractère mesuré du niveau d'indemnisation des administrateurs, au regard de leur implication. Un comité des rémunérations des dirigeants existe souvent déjà au sein des plus grands groupes coopératifs.

à la demande de la délégation sénatoriale à la prospective, sur les mobilités du futur. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

Quelques semaines plus tard, les « gilets jaunes » manifestaient pour protester contre les hausses de prix des carburants, qui grèvent le pouvoir d'achat de ceux qui n'ont pas de solution alternative à la voiture pour se déplacer. Nous sommes en train de vivre une révolution des mobilités, qui est très rapide : véhicules autonomes, véhicules électriques, véhicules partagés, applications de mobilité en temps réel, retour au vélo, nouveaux engins de déplacement personnel dans les villes, Pourquoi avons-nous choisi, avec le président de la délégation à la prospective, de nous intéresser à ce sujet ? Ce n'est pas seulement parce que c'est la mode ou pour recenser les dernières innovations technologiques plus seulement parce que se profilait la loi Mobilités. C'est, plus fondamentalement, pour cette raison évidente que la mobilité est l'une des conditions essentielles au développement d'un territoire dans toutes ses dimensions

Pendant près de cinquante ans, le développement de la mobilité se résumait à un seul type d'action : faire des routes, promouvoir la « bagnole » individuelle. Or, on le voit aujourd'hui, ce modèle trouve ses limites pollution, congestion, coût élevé au kilomètre des déplacements en automobile, dépendance économique au pétrole. Si la voiture a été un instrument de liberté formidable pour nos déplacements, on doit sortir du « tout-voiture », et c'est là que les difficultés commencent, notamment en raison du « tout-voiture solo Les transports collectifs, les transports partagés, le vélo en libre-service peuvent être mis en place dans les agglomérations, dans les zones denses, où les nouvelles technologies permettent d'enrichir l'offre de mobilités du quotidien. Mais comment faire dans les zones peu denses, dans les zones rurales où les start-up des mobilités ne viennent pas spontanément ? Les nouvelles mobilités connectées risquent de laisser sur le bord du chemin des pans entiers du territoire.

Actuellement, 80 % des espaces français métropolitains représentant 30 % de la population sont très mal, voire pas du tout desservis. Pour que le progrès technique dans le domaine des mobilités et les changements de pratiques en cours n'aggravent pas les fractures territoriales et ne créent pas une nouvelle fracture, une nouvelle frontière interne à notre pays, il ne faut pas être passifs et « attendre que ça se Bien au contraire, pour que le scénario positif des nouvelles mobilités au service de tous les territoires se réalise, il faudra un pilotage politique fort qui accompagne le progrès technique, qui l'encadre et qui l'organise. La mission confiée récemment à M. François Philizot sur la desserte fine des territoires va ainsi dans le bon sens. C'est à ce prix que la « mobilité augmentée » promise profitera à tous.

Avant, on testait, on imaginait des nouvelles solutions, on attendait éventuellement une réglementation, puis on voyait les nouvelles offres apparaître : le TGV a été longuement préparé ; la voiture a mis soixante ans pour se généraliser. Avec la nouvelle économie numérique, cela ne marche plus ainsi : des applications pour smartphones sont lancées, des vélos en libre-service sont déposés dans les rues des grandes villes- un peu n'importe comment -, des applications de réservation de voitures avec chauffeur concurrencent les bornes de taxi sans demander aucune autorisation à qui que ce soit.

celles-ci sont des politiques du temps long, avec des investissements lourds dans des infrastructures. Notre conviction est que l'innovation ne doit pas conduire à l'anarchie : nous réaffirmons donc qu'il est nécessaire qu'il existe un pilotage politique des mobilités à deux niveaux : celui des collectivités territoriales pour les mobilités de proximité, et celui de l'État pour la politique d'infrastructures

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur l'éminent président de la délégation à la prospective-

puisque les transports en France contribuent à hauteur de 30 % à nos émissions de gaz à effet de serre. Décarboner nos déplacements, cela paraît incontournable, et ce cap est désormais fixé avec l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2040. L'enjeu industriel est aussi fondamental. La chaîne de valeur se déplace, des constructeurs traditionnels vers les fournisseurs de services numériques, gestionnaires de données, ou encore fabricants de batteries, pour l'instant asiatiques ou américains. Une question se pose alors : va-t-on conserver une industrie des transports innovante en France et en Europe ? L'enjeu pour les finances n'est pas mince, avec près de 45 milliards d'euros de dépenses publiques. L'enjeu social est aussi prioritaire, l'absence de solution de mobilité frappant d'abord les plus vulnérables. Elle est facteur d'exclusion sociale et de frein à l'emploi, comme l'actualité en témoigne tous les jours. Les mobilités numériques posent également la question de l'exclusion numérique : l'illectronisme touche 6 à 11 millions de Français et il existe encore dans nos territoires ruraux des zones blanches.

Nous avons ensuite identifié trois critères qui influenceront les mobilités de demain. Premièrement, s'agissant des dynamiques territoriales des activités économiques et de l'habitat, va-t-on vers une polarisation accrue des territoires autour des métropoles et une spécialisation toujours plus forte des espaces ? Va-t-on, à l'inverse, vers une meilleure distribution des activités sur les territoires ? Deuxièmement, quel sera le coût des nouvelles mobilités et comment les financer ? Troisièmement, quels seront le degré d'intervention de la puissance publique et la coordination des acteurs ? Différentes combinaisons de ces critères dessinent des mobilités futures aux multiples visages : le pire, l'impensable serait le scénario des mobilités nouvelles pour les seuls territoires attractifs drainant les populations les plus favorisées. Une conviction forgée lors des auditions est que le progrès en la matière vient de micro-initiatives sur le territoire, qu'il s'agisse du covoiturage, de l'autopartage, du transport à la demande ou des pistes cyclables. Pour éviter de futures mobilités très excluantes, nous faisons donc plusieurs propositions. Première exigence : ces politiques doivent faire l'objet d'un pilotage à deux niveaux. Au niveau des collectivités- « agglo » et

suggérons de préserver une capacité nationale d'investissement dans les infrastructures de transport, assise sur des ressources pérennes, et de mettre en place des dispositifs de soutien aux actions locales en faveur des nouvelles mobilités, en particulier pour les territoires les plus défavorisés. deuxième exigence porte sur l'intermodalité. Nous préconisons de renforcer les alternatives à la voiture au-delà des coeurs d'agglomération, en veillant à assurer une desserte de qualité, en rapidité et en fréquence autour des zones denses et sur des plages horaires élargies,

Dernière exigence : ne pas subir des effets que nous n'aurions pas anticipés. Imposons l'ouverture des données mobiles, gardons sur notre territoire les start-up innovantes, encourageons l'expérimentation et captons les fonds européens de soutien à l'innovation. Nous préconisons enfin d'adapter l'action publique aux pratiques innovantes de mobilité, par exemple en permettant dans certains cas aux particuliers de participer à ces services. Parce que le progrès dans les mobilités, c'est aussi une nouvelle approche centrée sur les besoins des usagers, les débats à venir sur le projet de loi Mobilités seront l'occasion d'entrer plus dans

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la délégation à la prospective, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable aura très prochainement l'importante tâche d'examiner le projet de loi d'orientation des mobilités, qui a été déposé par le Gouvernement au Sénat le 26 novembre dernier. Nous sommes bien sûr déjà au travail et je suis honoré de la confiance que la commission m'a témoignée en me nommant rapporteur. C'est en cette qualité que je voudrais vous dire quelques mots en cette fin d'après-midi. J'en profite pour excuser notre président Hervé Maurey, qui n'a pas pu être parmi nous en cette fin d'après-midi en raison de la présence du Président de la République dans son département pour un autre débat, un peu plus vaste. Le thème de notre débat d'aujourd'hui- les mobilités du futur -est loin d'être sans lien avec les travaux que nous menons actuellement au sein de la commission. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'important travail de la délégation sénatoriale à la prospective ainsi que la qualité du rapport d'information qu'elle a publié en novembre dernier. Mais c'est aussi son rôle au sein de notre assemblée que je voudrais vanter. C'est en effet une grande chance pour nous de pouvoir compter sur les travaux de cette instance prospective qui, par nature, a le temps de se pencher et de réfléchir sur les défis du futur à 10, 15, 20 ans et au-delà, tandis que les commissions permanentes sont contraintes par les délais et les rythmes législatifs. Notre débat de cette fin d'après-midi, qui s'inscrit dans le contexte de l'examen très prochain du projet de loi d'orientation des mobilités, montre cette complémentarité. Quatre des cinq rapporteurs de la délégation sont d'ailleurs des membres actifs de notre commission et participent avec une grande assiduité aux auditions que je conduis et que j'ai souhaité ouvrir à tous les membres de la commission, en y associant également notre collègue Françoise Gatel, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je souhaite également les remercier pour leur travail, qui nous sera précieux lorsque nous arriverons à la phase concrète d'examen du projet de loi. Vous ne m'en voudrez donc pas de faire le lien, d'établir ce pont évident entre les réflexions prospectives de la délégation sur les nouvelles mobilités et le projet de loi d'orientation et de programmation que vous portez, madame la ministre, dans un contexte que l'actualité rend particulièrement sensible. Nous serions complètement déconnectés si nous nous contentions en cette fin d'après-midi de parler de la maturation technologique des véhicules autonomes ou encore des innovations scientifiques des start-up en matière de systèmes de covoiturage sans les relier aux enjeux actuels. Certes, les grandes mutations en cours doivent être bien comprises pour nous permettre de construire des scénarios d'adaptation à horizon 10 ou 15 ans. Mais ce sont surtout nos choix d'aujourd'hui que ces mutations bien appréhendées doivent déterminer. Le rapport de nos collègues identifie deux mutations principales, qui sont entremêlées. La première est une véritable « révolution » des usages. Cette révolution recouvre des enjeux environnementaux- comment passer à des transports moins polluants ? socio-économiques- comment garantir l'accès de tous à une offre de transport multiple et attractive ? -, industriels- comment permettre à notre filière automobile d'assurer les transitions en cours et à nos start-up de continuer à innover ? -, mais aussi territoriaux- comment mettre fin à ce qu'on appelle les « zones blanches de la mobilité », qui finalement qui finalement divisent les citoyens en deux catégories, les « connectés », reliés au monde extérieur et mobiles, et ceux qui ne le sont pas ? La seconde est une « révolution du numérique », qui impacte tant les offres de transports que la demande, tant les véhicules que les modes de conduite, et qui soulève des questions juridiques très fortes que le projet de loi d'orientation des mobilités commence à aborder. Ces questions sont très diverses. Elles vont de l'ouverture des données de mobilité au statut des personnes qui travaillent en ayant recours à des plateformes de mise en relation électronique. Notre monde change au gré de ces enjeux. Et, en tant que rapporteur de la LOM, mon principal message pour notre débat de cette fin d'après-midi sera d'insister sur la nécessité de penser les mobilités de demain comme un outil au service de la réduction des fractures qui parcourent notre société, au premier rang desquelles les fractures territoriales. Ainsi, nous devrons veiller à ce qu'il n'y ait pas des gagnants et des perdants dans cette révolution des mobilités. Nous devrons absolument faire en sorte que les mobilités du futur n'accentuent pas les inégalités existantes ou- pire ! -qu'elles La mobilité connectée, le covoiturage, les nouvelles offres de, le développement des transports à la demande ne doivent pas être réservés aux villes, tandis que les zones rurales n'auraient d'autre choix que de continuer à privilégier l'« autosolisme » et seraient même financièrement pénalisées pour cela, notamment en termes de fiscalité. Une très Une très récente étude du Pew Research Center montre que la spectaculaire progression des applis VTC aux États-Unis concerne avant tout les jeunes, les urbains et les catégories les plus aisées. Des mobilités du futur au service du désenclavement des territoires : voilà ce qui serait la plus grande des innovations ! Je rappelle d'ailleurs que c'est grâce à la présence des sénateurs au sein du Conseil d'orientation des infrastructures que les problématiques d'aménagement du territoire et du désenclavement des petites villes sont devenues des priorités. Et je souligne que cette présence est transpartisane. Le projet de loi d'orientation des mobilités comprend des dispositions dont l'ambition affichée est de répondre à ce sentiment d'abandon des territoires. On peut citer par exemple la couverture de l'ensemble du territoire par des autorités organisatrices de la mobilité, alors qu'aujourd'hui 80 % du territoire représentant 30 % de la population n'est pas couvert. On peut citer aussi la possibilité d'élaborer des plans de mobilité rurale, ainsi que l'ouverture des données de mobilité, qui doit permettre de faire connaître les solutions de mobilité dans les zones peu denses, ou encore la possibilité d'expérimenter des solutions de mobilité nouvelles dans ces mêmes zones. Quelques articles visent également à permettre le développement du covoiturage ou encore celui des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Mais seront-elles suffisantes ? Deux conditions me semblent essentielles. La première est celle d'un financement à la hauteur des enjeux, sincère et crédible. Beaucoup de solutions sont d'ores et déjà expérimentées par les territoires. Les initiatives doivent être soutenues, encouragées, développées. Les collectivités territoriales doivent avoir les moyens, les outils et les marges de manoeuvre nécessaires afin de pouvoir mettre en oeuvre ces solutions nouvelles. Tous les acteurs interrogés nous demandent de faire confiance à l'intelligence des territoires. C'est pour cette raison que le financement doit être transparent. Toutes les recettes perçues doivent être fléchées pour que les collectivités territoriales développent les offres de transport et créent des services partout, y compris dans les zones peu denses. La seconde condition en découle : les solutions de mobilité de demain doivent être construites en concertation avec l'ensemble des collectivités concernées. Les contrats opérationnels de mobilité conclus entre les autorités organisatrices et les régions, qui figuraient dans une version antérieure du projet de loi, étaient à mon sens de bons outils à l'échelle des bassins de mobilité. Voilà, mes chers collègues, le sentiment que je souhaitais vous livrer aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que les débats de cette fin d'après-midi alimenteront ceux que nous aurons très bientôt sur le projet de loi. En attendant, nos travaux continuent. Nous avons déjà mené plus de 65 auditions et elles se poursuivront durant tout le mois de janvier.

Monsieur le président, monsieur le président de la délégation à la prospective, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour ce débat sur les mobilités du futur et pour ce rapport d'information qui arrive au moment opportun pour éclairer le débat parlementaire que nous aurons prochainement sur le projet de loi d'orientation des mobilités. Les transports occupent une place centrale dans la vie quotidienne des Français, ils sont la condition nécessaire à l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé, à la culture et à de nombreux services. L'accès à la mobilité pour tous et partout est un facteur essentiel de la cohésion sociale et territoriale de notre pays. C'est la conviction forte que je porte et qui guide mon action. L'urgence environnementale nous oblige, par ailleurs, à prendre des mesures fortes pour réduire l'impact des transports sur l'environnement. La colère exprimée ces dernières semaines par les « gilets jaunes » montre l'importance de ce triple enjeu offrir à tous les Français l'accès à la mobilité, et que celle-ci soit à la fois abordable financièrement et soutenable pour l'environnement. Je crois profondément que les transformations que nous observons depuis plusieurs années dans les transports- révolution numérique ou émergence de l'économie du partage, par exemple -sont de réelles opportunités à saisir pour répondre à ces attentes. Elles offrent de nouvelles solutions de mobilité, alternatives à l'usage individuel de la voiture thermique, qui est encore trop souvent l'unique solution dans les territoires ruraux. Aussi, je partage les principaux constats du rapport d'information de votre délégation à la prospective, et je veux ici saluer la qualité du travail de vos rapporteurs. Le premier constat que vous faites, qui est au coeur du projet de loi d'orientation des mobilités, c'est celui de la nécessité d'apporter une solution de mobilité à tous et dans tous les territoires. Le projet de loi Mobilités, dont vous débattrez très prochainement, est la traduction de l'engagement du Président de la République de repenser en profondeur notre politique de mobilité en donnant la priorité aux déplacements du quotidien. Ce projet de loi a été nourri par un intense travail de concertation depuis les Assises nationales de la mobilité jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai la conviction que rien ne se fera en matière de transports sans un rôle actif et central des territoires, le premier pilier de ce projet de loi concerne la gouvernance des mobilités.

Cet objectif, que vous mettez en avant dans votre rapport, sera mis en oeuvre en privilégiant l'exercice de la compétence au niveau intercommunal et en faisant intervenir la région lorsque cela est nécessaire. Celle-ci sera cheffe de file de la mobilité sur son territoire. L'exercice de cette compétence mobilités sera simplifié, assoupli, et les collectivités se verront confier de nouveaux outils pour promouvoir des mobilités plus partagées et plus propres, en particulier à destination des publics les plus fragiles. L'exercice de ces compétences pourra s'appuyer sur le versement mobilité, l'actuel versement transport. La réflexion se poursuit avec les associations d'élus pour les situations où la collectivité ne souhaite pas organiser de transports réguliers. Je partage également l'orientation proposée par votre rapport de s'intéresser à des mécanismes pour les territoires où le potentiel fiscal du versement mobilité est inadapté aux besoins. Le deuxième pilier de cette loi est le soutien à l'innovation pour répondre aux besoins des territoires. C'est dans ce cadre que s'inscrivent la politique nationale d'ouverture des données de mobilité et le développement de services de billettique multimodale. L'objectif fixé dans la loi, et auquel nous travaillons avec les collectivités et les entreprises au sein du comité stratégique sur les données et la billettique multimodale, est simple il s'agit de favoriser le déploiement de nouvelles formes de mobilité en offrant à tous les Français, d'ici à la fin de 2021, toutes les informations sur la mobilité dans leur territoire. Cela répond notamment à votre proposition de construire des systèmes d'information des voyageurs de très haut niveau. C'est également dans ce cadre que s'inscrit la stratégie de la France en faveur du développement des véhicules autonomes, que j'ai présentée en mai 2018, avec une priorité donnée au développement des navettes autonomes. Le troisième pilier du projet de loi Mobilités vise à engager une transition complète de nos mobilités vers la neutralité carbone. Je crois profondément que cette transition ne sera possible qu'à travers de réels changements de comportement. J'ai la conviction que les mobilités actives, en particulier le vélo, peuvent jouer un rôle accru dans la mobilité des Français. C'est l'enjeu du plan Vélo, qui prévoit de tripler la part du vélo dans nos trajets quotidiens d'ici à 2024. le foisonnement créatif de ces nouvelles solutions ne doit pas nous faire oublier que, dans de nombreux territoires, la voiture restera le moyen de déplacement incontournable pour de nombreux trajets. L'enjeu, c'est donc de rendre les déplacements en voiture à la fois plus partagés, plus propres et plus économes. Je suis convaincue qu'en développant les mobilités actives et partagées, il sera ainsi possible à de nombreux ménages de se passer de leur deuxième, voire troisième véhicule. Aussi, le projet de loi prévoit de nouveaux outils pour inciter au partage des véhicules et a pour ambition de favoriser le déploiement de véhicules plus propres et plus économes. Le quatrième et dernier pilier du projet de loi Mobilités porte, pour les cinq prochaines années, sur un renforcement de l'investissement dans les infrastructures, avec une augmentation de 40 % par rapport au précédent quinquennat. Cet effort sans précédent ira en priorité aux infrastructures essentielles pour la mobilité quotidienne, avec notamment un grand plan de désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux. Là encore, et je sais que vous y êtes sensibles, c'est une révolution culturelle que nous entendons mener, où plutôt que de se contenter de promettre des grands projets, nous mettons notre énergie et nos moyens à ce qui sert vraiment le quotidien de nos concitoyens des routes et des voies ferrées en bon état, des trains là où il en manque, des itinéraires routiers enfin achevés. Au-delà de l'ensemble des mesures présentes dans le projet de loi Mobilités et des dispositions qui viendront l'enrichir lors des débats parlementaires, je sais que cette loi devra être accompagnée auprès de tous les acteurs pour qu'elle porte ses fruits. Les enjeux sont dans les territoires et sont donc aux mains de l'ensemble des porteurs de projet, collectivités, entreprises et associations. Vous en êtes sans doute les témoins dans chacun des territoires que vous représentez, comme je le constate moi-même à chacun de mes déplacements nos territoires regorgent d'initiatives et de solutions innovantes. C'est pour cela que j'ai lancé voilà maintenant un an la démarche baptisée French Mobility dans la continuité des Assises, pour créer un vrai lien de coopération et accompagner les porteurs de projet. Cette démarche facilite ainsi les expérimentations, fait partager les bonnes pratiques et accompagne les collectivités pour déployer des solutions de mobilité plus propres et plus accessibles partout sur notre territoire. Car c'est bien cela notre ambition commune : donner tous les outils, juridiques et opérationnels pour que les solutions concrètes se déploient. Vous l'aurez donc compris, les nouvelles mobilités, ce sont pour moi des mobilités qui incluent et rassemblent. Nous avons une responsabilité particulière pour nous assurer qu'elles n'oublient personne et qu'elles soient accessibles à tous et sur tous les territoires. Le grand débat qui débute est pour moi, pour nous tous, une nouvelle opportunité d'écouter les Français, de faire connaître nos actions. Vous le savez, nous avons choisi ensemble de décaler de quelques semaines le calendrier d'examen de ce projet de loi, pour tenir compte des propositions qui pourraient venir l'enrichir. C'est également le cas du débat d'aujourd'hui, avec vous, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, qui représentez nos territoires. Je vous remercie donc une nouvelle fois pour ce rapport et ce débat et je serai heureuse de répondre à vos questions. Nous allons pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

et c'est, par conséquent, réduire sensiblement la part du trafic routier, première cause de la pollution de l'air. De nombreuses villes souffrent de ce fléau et de la congestion automobile, qu'il est urgent de réguler. Pour répondre à cette problématique, l'avant-projet de loi d'orientation des mobilités autorisait initialement les grandes agglomérations à mettre en place des péages urbains. Si le principe majeur consistait alors à faire payer les usagers se rendant en centre-ville, ces mesures permettaient également de mettre en place un péage « inversé » ou « positif ». Cet « écobonus », tel qu'imaginé par la Métropole européenne de Lille ou encore la métropole de Grenoble, par exemple, prévoit de rétribuer les automobilistes volontaires qui évitent de prendre leur véhicule aux heures de pointe, utilisant un mode de transport plus doux ou optant pour le télétravail. Face aux revendications du mouvement des « gilets jaunes », qui dénonçaient, à juste titre, le risque d'un impôt injuste pénalisant les ruraux et ceux qui ne peuvent habiter plus près de leur lieu de travail, le Gouvernement a intégralement supprimé du projet de loi final les articles relatifs aux péages urbains, sans se douter que les deux systèmes- l'un qui pénalise et l'autre qui récompense les conducteurs -étaient liés dans le texte. Faute de cadre juridique, il est aujourd'hui impossible de lancer l'expérimentation de ces péages inversés. Aussi, je vous demande, madame la ministre, ce que le Gouvernement entend faire pour que le projet de loi évolue afin de permettre ces expérimentations.

avaient pour objectif de mieux encadrer celui-ci. Or il est apparu que cette disposition était mal comprise et il nous a donc semblé préférable de la retirer du projet de loi. S'agissant du péage « inversé » ou « positif » tel que l'envisage la Métropole européenne de Lille, et comme vous l'avez évoqué, il s'agit, grâce à un ciblage des usagers fréquents concernés, de récompenser ceux qui renoncent à des trajets aux heures de pointe sur les axes urbains les plus encombrés. Effectivement, l'expérience montre qu'avec un report d'une fraction finalement assez limitée de ces usagers, on peut réduire significativement la congestion. Le projet de péage « inversé » a emporté l'adhésion, depuis 2017, des services de l'État, mais il apparaît que tel qu'il est envisagé aujourd'hui, il supposerait un recours large, pour le ciblage en amont des usagers, à des moyens de vidéosurveillance et au croisement du fichier des immatriculations pour enregistrer les comportements. Cela peut représenter une atteinte à la vie privée disproportionnée compte tenu de notre cadre constitutionnel. Or c'est un point de vigilance du Gouvernement : toutes les dispositions du projet de loi d'orientation des mobilités liées aux dispositifs de contrôle automatisé ont fait l'objet d'une analyse rigoureuse quant à leur proportionnalité.

Une catastrophe sanitaire se prépare. D'une manière plus générale, il faut absolument entendre et accompagner les collectivités territoriales et les métropoles, qui ont des capacités à innover.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en dépit de l'issue en demi-teinte de la dernière COP, la lutte contre le réchauffement climatique est devenue un impératif. Parmi les énergies nouvelles, il en est une qui me semble particulièrement sous-employée, à savoir l'hydrogène, qui, en production totalement décarbonée, n'émet aucune pollution et qui, utilisé comme carburant, permet alors le recours à des véhicules électriques, moyennant une énergie totalement propre, même si elle reste un peu coûteuse. Les technologies développées aujourd'hui le rendent adaptable aux transports individuels comme aux transports collectifs et déclinable sur tout type de véhicule. Certes, notre pays vient de se doter d'un plan national hydrogène. C'est une première, une étape importante qu'il convient de souligner. Mais il faut être plus ambitieux : il me semble nécessaire d'assurer rapidement le développement d'une filière française performante, compétitive et innovante. Trop souvent, notre pays a souffert du retard pris sur ses voisins : j'en veux pour exemple la signature par Alstom de plusieurs contrats avec les dans le domaine du ferroviaire, que la France ne sortira son premier train à hydrogène qu'en 2022. Les études établissent aujourd'hui que d'ici à 2040, les véhicules à hydrogène constitueront seulement le quart des véhicules circulant.

dès cette année pour accompagner l'émergence de cette filière afin qu'elle joue un rôle central dans notre transition écologique. En particulier, dans quelle mesure les collectivités seront-elles incitées pour leurs propres flottes de transport, mais aussi pour leurs services de transport collectif et leur développement économique, à recourir à l'hydrogène ? l'AFHYPAC, qui regroupe les acteurs de la filière, annonce des possibilités d'exportation d'un hydrogène produit en France à hauteur d'environ 6 milliards d'euros d'ici à 2030. Là encore, quelles actions le Gouvernement entend-il mener pour ne pas passer à côté de telles opportunités de développement ? La parole Monsieur le sénateur, je peux vous assurer que le Gouvernement est convaincu que l'hydrogène a un rôle important à jouer dans la transition énergétique. une solution de mobilité propre complémentaire au bio-GNV et aux batteries et c'est également un vecteur de décarbonation du réseau gaz. La filière française est en avance et compte de nombreux industriels de premier rang mondial, présents sur toute la chaîne de valeur. Le plan de déploiement de l'hydrogène, qui a été présenté le 1 juin dernier, veut capitaliser sur ces atouts pour développer les avantages industriels français

en particulier pour les véhicules lourds, les poids lourds, les véhicules utilitaires ou les trains, et pour les flottes captives. Le plan comporte plusieurs dispositions opérationnelles. Tout d'abord, les dispositifs de soutien au verdissement des véhicules ont été systématiquement élargis à l'hydrogène je pense au suramortissement pour les poids lourds ou à celui qui a été introduit pour les navires, au bonus pour l'acquisition de nouveaux véhicules ou à la prime à la conversion. Deuxième dispositif : le soutien à l'émergence d'écosystèmes, qui a fait l'objet d'un appel à projets spécifique de l'ADEME- écosystème de mobilité hydrogène. Il s'agit non seulement de développer des solutions de mobilité, mais aussi de disposer de systèmes de production d'hydrogène. L'appel à projets, lancé en

sur le développement du train à hydrogène, mission conduite par le député Benoît Simian et qui doit nous permettre de déployer une expérimentation de trains à hydrogène avant la fin du quinquennat. L'hydrogène, je vous le confirme, est un vecteur important pour les mobilités. C'est même le cas pour le vélo puisque l'entreprise Pragma Industries a été récompensée au Consumer Electronic Show de Las Vegas cette année pour son vélo à assistance électrique à hydrogène.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de multiples facteurs favorisent et même imposent l'émergence de nouveaux modes de mobilité. L'usage du véhicule individuel à énergie fossile va sortir de nos pratiques quotidiennes. Les territoires les plus urbanisés sont pour la plupart organisés avec des solutions alternatives de transport collectif. La situation est bien différente en milieu rural, où, pourtant, le fait de pouvoir se déplacer sur des distances parfois longues est un impératif incontournable du quotidien. Face à l'obligation du changement, de nombreuses propositions techniques émergent, qui font intervenir autant des start-up que des grandes entreprises des secteurs traditionnels. Comme l'expose l'excellent rapport d'information produit récemment par nos collègues et amis de la délégation à la prospective, le cadre institutionnel des mobilités est bousculé par toutes ces innovations. Il se pose des questions pratiques de partage de l'espace public, entre piétons, cyclistes, utilisateurs de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel ». Se posent également des questions de responsabilité assurantielle. En imaginant que les choses, comme toujours, iront plus vite qu'on ne l'imagine, je me pose la question de la cohabitation des différents types de véhicules pendant quelques années. Comment gérer sur une même voie des véhicules parfaitement autonomes et d'autres qui ne le seraient absolument pas ? La question de la relation directe entre chauffeurs, avec le cortège de coups de klaxon et de noms fleuris qui les accompagne, ne sera sans doute un problème que pour quelques-uns- j'espère un épiphénomène. Au-delà de la boutade, il y a un vrai problème, et c'est l'objet de ma question madame la ministre, les véhicules des deux générations évolueront-ils sur des voies dédiées différentes ? Sinon, quelles solutions sont à l'étude ? Avez-vous envisagé, dans les années qui viennent, des mesures pour que la cohabitation se mette en place progressivement sans doute, prioritairement en milieu de circulation peu dense, à savoir en milieu rural, ce qui serait probablement plus sécurisant et donnerait des perspectives à des territoires où les solutions de mobilité sont essentielles ? La parole est à Mme la ministre. est à Mme la ministre. La question de la cohabitation des véhicules autonomes avec les autres véhicules est un enjeu essentiel en termes d'innovation, mais aussi d'acceptabilité. D'ores et déjà coexistent, à la fois sur le marché et sur nos routes, des véhicules qui disposent d'assistant de conduite, notamment l'adaptation automatisée de la vitesse, le maintien sur voie, le freinage d'urgence automatisé. Ces dispositifs ont précisément vocation à gérer les interactions avec le trafic dans un sens qui améliore la sécurité routière. Les futurs systèmes autonomes devront aussi gérer la complexité des interactions avec les autres usagers, qu'il s'agisse des autres automobilistes, mais aussi des vélos et des piétons, et des piétons, et ce en toute sécurité. Cela fait partie des expérimentations qui sont soutenues par l'État dans le cadre de la stratégie pour le développement des véhicules autonomes. Ces expérimentations doivent notamment nous permettre d'améliorer les connaissances sur les conditions d'acceptabilité de ces véhicules. C'est un point essentiel du cadre de validation de ces systèmes que nous sommes en train de construire avec les acteurs. S'agissant des transports publics autonomes et notamment des navettes, je partage tout à fait le souci qu'ils puissent bénéficier à tous les territoires, y compris les territoires ruraux. C'est une priorité de notre stratégie sur le véhicule autonome. Je suis convaincue que ce sont les collectivités, lesquelles connaissent à la fois les besoins et les conditions de circulation et de sécurité, qui sont les mieux placées pour porter des projets de navettes autonomes. Les expérimentations déjà soutenues par l'État et celles qui sont sur le point de l'être dans le cadre d'un appel à projets en cours ont permis de faire remonter des cas d'usage variés, notamment en en milieu rural, et je m'en félicite. L'État poursuivra son soutien aux projets innovants en milieu rural, dans le cadre des appels à projets, mais aussi dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. J'invite tous les porteurs de projets à se saisir de ces outils. Je demande

Monsieur le président, monsieur le président de la délégation, madame la ministre, mes chers collègues, l'actualité le montre chaque jour : la mobilité est un enjeu essentiel pour les Français, dans leur quotidien, pour leurs trajets personnels et professionnels. Nous le constatons depuis longtemps : nous sommes arrivés à un point de rupture- une rupture technologique -dans les besoins des usagers, dans le coût de la mobilité. Il convient d'accompagner au mieux les citoyens et les territoires dans cette transition pour qu'elle soit une chance pour tous, il faut veiller à préserver la liberté de circuler de chacun. Les mobilités nouvelles doivent donc être faciles, accessibles, rapides et peu coûteuses. Tout à par le développement de nouvelles technologies innovantes, par l'amélioration des infrastructures, par la mise en place d'incitatifs financiers pertinents. La mobilité du futur doit être plurielle, intelligente collaborative, propre, solidaire et responsable. Quel programme ! La mise en place d'un cadre réglementaire fort et incitatif doit permettre de sortir de la dépendance à la voiture, d'accélérer la croissance des nouvelles mobilités tout en prenant en compte la diversité et la spécificité de nos territoires ruraux. Dès lors, madame la ministre- je sais quelle est votre détermination comment faire en sorte que les mobilités du futur, toutes plus innovantes les unes que les autres, soient adaptées tant au milieu urbain qu'au milieu rural- et j'insiste -, en veillant à respecter leur diversité et leurs spécificités ? Comment utiliser ces mobilités innovantes pour reconnecter le rural et l'urbain ? La parole est à Mme la ministre. est à Mme la ministre. Je partage tout à fait votre préoccupation. L'enjeu est de faire en sorte que la révolution des mobilités puisse être mise à profit pour améliorer concrètement la mobilité de tous nos concitoyens, qu'ils résident ou travaillent en milieux urbains, ruraux ou périurbains. L'innovation en particulier ne doit pas être un privilège réservé aux citadins ; elle doit au contraire profiter à tous et partout. Nous avons dans nos territoires des collectivités, des entreprises, des associations, des citoyens qui portent des solutions innovantes pour améliorer les déplacements du quotidien et il nous faut les soutenir. C'est pour cela que j'ai lancé voilà maintenant un an la démarche d'appel à projets French Mobility, qui a pour ambition de soutenir l'expérimentation, le développement et la diffusion dans tous les territoires de toutes les innovations au service de la mobilité du quotidien. projets innovants de mobilité en territoires ruraux et périurbains sont par exemple soutenus en ingénierie pour couvrir des thématiques aussi variées que le déploiement de mobilité active et partagée, le soutien à l'intermodalité en milieu rural, le déploiement de services de mobilité pour des publics spécifiques, la mise en oeuvre de systèmes autonomes. Je vais poursuivre cette dynamique et autant de territoires seront sélectionnés dans les prochaines semaines. Afin de partager ce qui marche dans les territoires, une plateforme rendant visibles tous ces projets sera mise en place à très brève échéance. Par ailleurs, afin que l'ensemble de nos concitoyens sachent quelles sont les solutions de mobilité qui se trouvent à leur proximité, les régions seront chargées de s'assurer que, d'ici à 2021, l'ensemble de leurs territoires soient couverts par un système d'information numérique sur les solutions de mobilité qui existent. La parole me satisfait pleinement. est à M. le rapporteur. Madame la ministre, cette question de la mobilité, notamment dans les territoires ruraux et périurbains, infuse le débat qui parcourt aujourd'hui notre société. On l'a vu cet après-midi dans l'échange entre le Président de la République et les maires : ce sujet a été posé à de nombreuses reprises. La réponse à cette question de « comment mieux se déplacer, à moindre coût », dans des territoires où la voiture individuelle n'a pas d'alternative, constitue une des solutions à mettre en oeuvre pour résorber cette crise. mobilités, ou LOM, sera l'occasion de débattre sur ces choix, mais je souhaitais aujourd'hui vous apporter une illustration de ce qu'il est possible d'imaginer, de l'intelligence que nos territoires peuvent mobiliser pour trouver des solutions innovantes.

Le constat a été fait de ces phénomènes d'étalement urbain, depuis plusieurs dizaines d'années, conduisant à une mobilité de plus en plus éclatée et logiquement à l'utilisation croissante de la voiture. Ce constat est indéniable. Il faut ajouter à cela que nos concitoyens ne comprennent pas toujours les limites administratives de leur bassin de vie. Ils ne comprennent pas, par exemple, pourquoi un bus ne va pas un peu plus loin parce qu'il n'est plus dans le même territoire. On le voit, l'innovation, l'intelligence territoriale peut largement contribuer à la vie de nos concitoyens dans leur demande de mobilité. l'exemple du sud-Isère mérite d'être reproduit largement. Mais je crois aussi qu'il faut aller au-delà et permettre notamment aux territoires périphériques de constituer avec leurs voisins des communautés de projets au service des mobilités. Ces territoires n'ont bien souvent aujourd'hui pas la taille critique, l'ingénierie, la cohérence géographique, les finances pour organiser les mobilités. Mais ils pourraient, avec leurs voisins plus importants, créer la communauté que j'évoque. Des freins peuvent exister, réglementaires ou législatifs notamment on pense par exemple au versement transport, dont le taux unique sur un vaste bassin peut être un obstacle. Je crois important de pouvoir identifier ces freins et les lever dans le cadre de nos futurs débats pour faire en sorte que l'exemple dont je parlais puisse être reproduit et élargi. J'aimerais donc connaître, madame la ministre, votre positionnement sur cette question. Il faut conclure, monsieur le rapporteur. Comment favoriser des projets de coopération au service de nos concitoyens ? La parole est à Mme la ministre. est à Mme la ministre. Je suis convaincue que c'est effectivement par une bonne coopération entre les différentes collectivités que l'on pourra développer des offres de qualité à l'échelle de bassins de mobilité, qu'ils soient urbains ou ruraux. C'est, de ce fait, une ambition forte du projet de loi d'orientation des mobilités. Ainsi, celui-ci prévoit une meilleure coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité et, plus largement, les acteurs de la mobilité à l'échelle de ces bassins de mobilité. Les régions et les autorités organisatrices de la mobilité auront à se coordonner et à définir les modalités de leur action commune, par exemple au travers d'un contrat opérationnel de mobilité. Le terme n'est plus employé dans le projet de loi, mais je pense qu'il pourrait effectivement y être réintroduit. C'est une des modalités de cette coopération, qui doit permettre à la fois d'assurer la cohérence, la complémentarité des différentes formes de mobilité, l'intermodalité en termes de dessertes, de tarification, d'horaires, d'information, d'accueil du public, la création et l'aménagement de pôles d'échanges multimodaux

aussi le rapprochement dans des syndicats mixtes particuliers des différentes autorités organisatrices, en permettant de moduler le taux du versement mobilité- ce qui est aujourd'hui impossible -au sein d'un syndicat mixte,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme un préalable à l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités, qui a été repoussé, nous entamons cette nouvelle année par un débat sur les mobilités du futur. Ma question, et j'en suis désolée, se fera un peu provocatrice. Si nous encourageons évidemment le développement de nouvelles mobilités, qu'elles soient actives ou autonomes, nous estimons que la question du transport collectif de masse, c'est-à-dire le transport ferroviaire, doit rester la pierre angulaire de toute politique publique des transports, et ce y compris au regard des enjeux climatiques, le rail étant un mode bien moins polluant que la route et un puissant levier pour lutter contre la désertification rurale. Pourtant, les petites lignes ne cessent de fermer, de petites gares sont supprimées et on limite l'offre notamment des trains de nuit. Aujourd'hui, on demande même aux postiers de jouer les chefs de gare Nous sommes donc aujourd'hui très loin des 62 000 kilomètres de rails des années 1930 puisque le réseau ferroviaire a été divisé par deux. Le rapport Spinetta, conjugué à la funeste réforme ferroviaire, promet pour bientôt la suppression de 10 000 kilomètres de lignes capillaires jugées trop peu rentables, les usagers étant appelés à se réorienter vers les bus, l'autopartage, le vélo ou toute autre mobilité

que quand on passe du car au train, on en gagne 65 % ». Madame la ministre, allez-vous préserver ces lignes et ces infrastructures comme autant d'outils pour lutter contre le dérèglement climatique, qui est l'affaire du siècle ? Et pour l'aménagement des territoires, allez-vous enfin considérer le ferroviaire non pas comme une mobilité du passé, mais bien comme une mobilité d'avenir ? Très bien ! La parole

d'une augmentation de 50 % des moyens consacrés à l'entretien et à la régénération du réseau ferroviaire. Notre programmation des investissements, celle qui figure dans le projet de loi d'orientation des mobilités, dont vous aurez prochainement à débattre, prévoit aussi le développement du transport ferroviaire, notamment pour avoir de véritables RER métropolitains autour des métropoles régionales, évidemment de continuer à moderniser le réseau en Île-de-France. Je me réjouis de voir que les présidents de région et les présidents de métropole se saisissent de ces sujets. Il ne s'agit pas d'oublier les lignes de desserte fine des territoires. Je viens de confier une mission au préfet François Philizot afin de travailler avec chacune des régions à partir des solutions techniques qui ont été identifiées à ma demande par SNCF Réseau pour réfléchir à des modalités

quelques trains par jour- jusqu'à un ou deux trains. Il faut non seulement réfléchir à l'adaptation des solutions techniques, mais aussi trouver les bonnes organisations pour gérer au mieux ce réseau de desserte fine des territoires

de ramener des voyageurs et d'assurer leurs correspondances. Je suis convaincue qu'elles seront aussi un outil pour favoriser le redéveloppement, la relance du transport ferroviaire dans nos territoires.

Mme la présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, avec Mme la maire de Paris, Anne Hidalgo, a remis en cause la liaison Charles-de-Gaulle Express

inscrits dans un contrat de plan État-région qui a vocation à traduire une volonté commune, comme son nom l'indique, de l'État et de la région. Je voudrais souligner que le contrat de plan État-région en Île-de-France n'a pas été modifié depuis l'arrivée de notre gouvernement, faute de demande émanant de la région : nous mettons donc en oeuvre le contrat de plan tel qu'il avait été signé par nos prédécesseurs. Je voudrais également souligner que, contrairement à ce qui a cours dans les autres régions,

l'État a préféré accorder un prêt du Trésor ; il n'y a pas un euro de subvention publique, et cela restera le cas tout au long du projet. Je vais évidemment prendre en compte les avis des collectivités. Je prends également en compte l'enjeu national que représente la plateforme Charles-de-Gaulle, qui est notre premier national. J'écouterai Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, tout en notant que l'une et l'autre ne disent pas la même chose, voir disent le contraire. Nous mènerons donc ce projet

Mais l'actualité chez nos voisins britanniques doit nous amener à connaître ce soir, par un vote qui doit intervenir à la chambre des représentants, la position de la Grande-Bretagne sur les modalités du Brexit. Or il se trouve que, sans même attendre de connaître l'issue de ce vote, par la voix de Chris Grayling, ministre du gouvernement de Mme May, nous apprenons la décision de mettre sur la table 100 millions de livres à partager entre trois opérateurs, Brittany Ferries, DFDS et Seaborne Freight, afin de soutenir l'ouverture de nouvelles lignes sans passer par Douvres et, par conséquent, sans passer par Calais. Vous comprendrez dès lors que je profite de votre présence aujourd'hui au Sénat pour vous dire l'émoi que suscite une telle annonce, à quelques semaines du 29 mars. Je ne rappellerai pas ici ici par quoi sont passés les opérateurs du port de Calais et l'ensemble des acteurs économiques tout comme ceux du tunnel ces dernières années. Il est par ailleurs choquant de voir que nos voisins et amis britanniques

sur les procédures de contrôles et, surtout, sur les délais de celles-ci ? Enfin, un tel soutien à ces trois entreprises vous semble-t-il répondre aux règles en vigueur en matière de libre concurrence ? La parole est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, j'ai bien eu connaissance de l'initiative du gouvernement britannique de réserver des capacités chez un certain nombre d'armateurs, pour faire face à l'éventualité d'une congestion des trafics sur les ports existants. Nous avons effectivement demandé des explications au gouvernement britannique- je ne suis pas en mesure de vous les donner aujourd'hui -à la fois sur la procédure

Nous y travaillons depuis ces derniers mois, notamment pour renforcer les moyens permettant de réaliser les contrôles douaniers et sanitaires

pour disposer d'espaces propres à ces contrôles. Vous le savez, des financements ont été réservés au niveau du mécanisme d'interconnexion européen européen pour les ports du réseau global. En outre, un nouvel appel à projets sera lancé l'an prochain pour les ports du réseau central dont fait partie Calais, qui, dans ce cadre, peut donc bénéficier de taux de subvention importants. pour accélérer la réalisation de ces aménagements et prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la continuité, notamment, des services de transport,

On peut par exemple s'interroger sur la place qui sera laissée aux nouveaux engins de déplacement- trottinettes, gyropodes et autres hoverboards -en milieu urbain. Faudra-t-il leur consacrer des voies spécifiques, faudra-t-il les intégrer dans les futurs plans de circulation des villes ? L'État contribuera-t-il aux dépenses ainsi engendrées ? De manière générale, la stratégie de l'État en faveur des transports de demain aura-t-elle comme priorité de développer les nouvelles mobilités urbaines ou s'attachera-t-elle à résorber d'abord les carences en milieu rural ?

Vous avez parlé, madame la ministre, d'un effort de l'État majoré de 40 % sur le ferroviaire et le routier. Pouvez-vous nous donner des précisions quant à sa répartition ? De plus, le rapport sur les nouvelles mobilités, fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective, préconise la mise en place de mécanismes de soutien aux actions locales pour les territoires enclavés. Vous avez lancé en 2018 un appel à manifestation d'intérêt sous le nom de French Mobility. La date limite de dépôt des candidatures était fixée à la fin octobre 2018. Avez-vous reçu des propositions et des solutions particulièrement pertinentes qui pourraient faire l'objet d'expérimentations à court terme, voire d'une mise en oeuvre plus globale sur l'ensemble des territoires concernés ? La parole

mais en partant du constat que, spontanément, les offres innovantes en termes de mobilité ont tendance à se concentrer dans les grandes villes : toutes les start-up ont envie de montrer ce qu'elles savent faire à Paris, à Toulouse Le rôle de la puissance publique, c'est bien que cette innovation profite à tous les territoires. Le coeur de la politique en termes de programmation des infrastructures sera en priorité, je le redis, l'entretien, la régénération des réseaux routiers et ferroviaires et un plan de désenclavement routier avec l'accélération de projets qui sont souvent promis depuis des décennies-

les collectivités pour sortir des zones blanches de la mobilité et pour apporter des solutions alternatives à l'usage individuel de la voiture dans tous les territoires. Cela passe d'abord par le fait de faciliter l'exercice de la compétence par les collectivités, comme le prévoit le projet de loi d'orientation des mobilités. Cela passe ensuite, on l'a évoqué, par le fait de permettre aux petites intercommunalités de travailler avec les plus grosses, à travers une modulation du versement transport, demain du « versement mobilité

il serait heureux d'introduire une cohérence, peut-être au travers des futurs CPER, et que l'État sache aussi accompagner, en matière d'infrastructures et de mobilité, le soutien à ces filières et aux emplois qu'elles représentent. La

De façon générale, quand on parle de mobilités, nous sommes sur des compétences décentralisées, et il ne s'agit donc en aucun cas, de la part de l'État, de vouloir faire à la place des collectivités. L'État porte des infrastructures de transport

du bloc communal et au niveau régional. Cette architecture me semble la bonne sur l'ensemble de notre territoire. C'est pourquoi nous allons oeuvrer, au travers de la loi d'orientation des mobilités, pour que, justement, cette compétence soit exercée par l'ensemble des intercommunalités, le cas échéant regroupées en bassins de mobilité dans le cadre de syndicats. Cela permettra, le cas échéant, une mutualisation des ressources, avec la région

exercée par les intercommunalités de la région à la fois sur les déplacements d'intérêt régional et sur la cohérence, la coordination est la bonne. S'agissant de la situation en Île-de-France, l'État ne s'en mêle pas davantage : c'est Île-de-France mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France,

Mme Victoire Jasmin. Madame la ministre, mes chers collègues, je tiens au préalable à féliciter la délégation sénatoriale à la prospective pour la qualité de son travail. Ce débat est une opportunité qui me permet d'évoquer la problématique du transport dans les territoires d'outre-mer. En effet, en matière économique, environnementale, mais aussi en termes d'équité territoriale et sociale, il est urgent pour nos territoires et plus singulièrement pour la Guadeloupe, qui est un archipel, d'organiser un service public des mobilités afin d'assurer la la continuité territoriale de façon optimale et satisfaisante pour l'ensemble de la population. Ainsi, une autorité de régulation unique, dont la gouvernance serait collégiale entre l'État, les collectivités locales et les prestataires privés, pourrait gérer de façon mutualisée tous les modes de déplacements individuels ou collectifs, de passagers ou de marchandises, maritime, routier et aérien, à l'échelle de l'ensemble de l'archipel. L'objectif est, grâce à une péréquation horizontale des dessertes les plus efficientes vers les zones les plus enclavées, de permettre un égal accès à tous à un service public intégré, multimodal, régulier et de qualité. Cela aurait de décongestionner les axes routiers déjà saturés, dont l'impact nocif sur la qualité de l'air est avéré, tout en permettant de rationaliser le financement des investissements structurants, la maintenance des infrastructures, ainsi que la formation des personnels et la sécurité des usagers.

depuis que le seul bateau qui assurait la desserte vers l'île a cassé son moteur. Seuls les marins-pêcheurs acceptent d'assurer les déplacements des usagers, ce qui reste une alternative précaire en attendant une solution palliative sécurisée et respectueuse de la législation en vigueur.

au coeur de mes préoccupations. Je suis convaincue que, à la Guadeloupe comme dans les autres régions, il est effectivement très important d'assurer une prise de compétence, et que, sur l'ensemble du territoire, les collectivités s'organisent pour proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle qui permettent de lutter contre la congestion et la pollution.

Peut-être serait-il intéressant de creuser aussi l'hypothèse, émise dans certaines régions, d'un syndicat, ce qui permettrait de regrouper à la fois le niveau intercommunal, les différentes autorités organisatrices

En tout cas, je suis certaine que l'on peut, et que l'on doit progresser pour offrir des solutions alternatives, y compris en prenant en compte les enjeux de sécurité routière que vous avez mentionnés, les

là encore, des compétences des collectivités locales. Mais je peux vous assurer que le préfet a mobilisé les services de l'État pour regarder comment on peut appuyer techniquement l'émergence de solutions, sans attendre la réparation du navire actuellement indisponible. La parole

De nombreux maires ont parlé de cette fracture en matière non seulement d'enclavement, qu'il soit numérique, ferroviaire ou routier, mais également de mobilité, puisque, vous le savez, dans les territoires les plus ruraux, il est plutôt difficile de mettre en place des transports en commun. Madame la ministre, ma question va être simple. L'heure n'est plus au constat,

voire d'une troisième voiture. C'est vraiment tout le sens de la loi d'orientation des mobilités de permettre aux collectivités de se saisir de cet enjeu, de les accompagner, de déployer les solutions innovantes, précisément pour répondre à ces territoires et à nos concitoyens qui se sentent abandonnés.

À la suite des travaux du Grenelle de l'environnement, en juillet 2010, a été inscrit dans la loi l'objectif d'une division par quatre des émissions sur le territoire national. Les véhicules électriques présentent un énorme avantage pour atteindre cet objectif

Comme en matière d'énergie solaire, il me semble important de considérer le cycle de vie de ces véhicules, et en particulier de leur batterie, dont la durée de vie est estimée à dix ans.

Or le lithium métallique réagit avec l'azote, l'oxygène et la vapeur d'eau dans l'air. De plus, l'hydroxyde de lithium présente un risque potentiel significatif, car il s'agit d'un composé extrêmement corrosif qui peut s'avérer nocif, notamment pour les organismes aquatiques. le recyclage des batteries est une condition indispensable au succès écologique des véhicules électriques. Aujourd'hui, des efforts sont faits, en particulier au travers des investissements d'avenir, dans le domaine de la recherche et du développement. Mais la filière du recyclage sera-t-elle prête lorsque les premiers volumes de batteries arriveront en fin de vie ?

les émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez, nous nous sommes fixé pour objectif de multiplier par cinq le nombre de véhicules électriques vendus en France d'ici à la fin du quinquennat. Nous avons également plaidé en faveur d'objectifs ambitieux à l'échelle européenne,

faisons en sorte que les nouvelles mobilités soient aussi une avancée pour eux et non un énième instrument de relégation, de frustration, et donc de colère. Les 80 kilomètres à l'heure ont pénalisé les territoires. Il est vécu comme punitif. Il a été et il est l'un des détonateurs du mouvement des « gilets jaunes ». Or de nombreux territoires ont besoin de moyens et de considération afin que les nouvelles mobilités soient aussi une chance pour eux.

L'ensemble de ces mesures commencent à produire leurs effets. Je vous invite notamment à vous reporter aux données publiées récemment par l'ARCEP : ce plan de couverture numérique est bien en train de se déployer.

durable. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la délégation à la prospective, mes

Notre délégation à la prospective est donc bien à sa place en inscrivant précisément ses travaux dans cette temporalité. Nous devons avoir une vision claire de la manière de déployer les nouvelles mobilités dans tous les territoires. Nous devons également comprendre les grands enjeux et les objectifs liés aux mobilités,

convient de poser la question délicate du financement des transports. Cette problématique ne disparaîtra pas par enchantement dans le futur, tant s'en faut, d'autant que les différents modes de transport ont des clefs de financement très différentes. Les grandes infrastructures resteront à la charge de la collectivité publique

du système français, fondé sur le versement transport, qui est un financement solidaire, n'est pas remise en cause à ce jour. Mais un nouveau débat sur la fiscalité écologique et la taxation ou mise à contribution des externalités négatives doit être rapidement pas une remarque, mais une série d'interrogations. La pratique du partage et le paiement à l'usage vont-ils se généraliser ? La location de la trottinette, du vélo ou de la voiture va-t-elle supplanter le modèle d'achat et de propriété qui est le nôtre Les expériences de mutualisation fonctionnent bien, parce qu'elles permettent aux usagers de faire des économies en optimisant leurs coûts ; et, grâce à des plateformes numériques très accessibles, les différents acteurs peuvent se mettre en relation de manière simple.

Nous ne pensons pas que les zones peu denses soient condamnées à être les grandes oubliées des mobilités du futur. En la matière, les obstacles sont largement surmontables, et nos propositions vont précisément dans dans ce sens. C'est forts de cette conviction que nous affirmons que les mobilités du futur peuvent être inclusives en s'adressant à tous. Les nouvelles technologies peuvent même nous aider à favoriser ce caractère inclusif. L'ensemble de ces remarques et questionnements seront au coeur de nos réflexions relatives au projet

du mardi 15 janvier 2019, un vote favorable, d'une part, à la nomination de M. Jean Cabannes- 27 voix pour, 2 voix contre -et, d'autre part, à celle de Mme Natalie Fricero- 29 voix pour, aucune voix contre -aux fonctions de membre du Conseil supérieur de la magistrature.